la parole est à notre collègue Gilbert Roger. et l'ajournement d'étudiants au concours de la fonction publique territoriale. Des témoignages de plus en plus nombreux parviennent d'étudiants refusés au concours de la fonction publique avec une note proche de celle qui est nécessaire. Ces derniers, le plus souvent sont laissés pour compte par exemple je connais le cas d'une jeune étudiante ajourné à l'agrégation pour seulement 1. Aucune proposition ne lui a été faite. Or ces secteurs doivent remédier aux démissions manque d'intérêt dans la profession, les rectorats se voit même obligé de trouver des contractuelles en speed dating, comme l'ont dit et de les former en quelques jours. Un métier complexe quelles mesures pourraient être prises immédiatement par le gouvernement prendre contact avec les ajourner leur proposer des postes de contractuels avec pour échéance la titularisation. Merci. Merci, cher collègue, la parole à Madame la Ministre Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et la formation professionnelle. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Gilbert Roger effectivement chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste principale que par ordre de mérite. Les candidats aptes au jury. Si la liste principale et complète le juré peut établir une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne pourrait pas être nommé l'appréciation, je le rappelle de la qualité des prestations des candidats à un concours relève de la compétence souveraine des jurys. Et ces décisions ne sont pas susceptibles de recours devant les juridictions administratives dès lors que les jurys ont fonctionné et délibérée de manière régulière. Hormis le le cas très spécifiques du recrutement par la voie contractuelle de personnes en situation de handicap qui donne lieu à la titularisation à l'issue du contrat aucune disposition législative ne permet actuellement de recruter un agent contractuel au sein de la fonction publique et de titularisés sans concours. La baisse du nombre de candidats. Enregistrés au concours de recrutement de professeurs du 1er et second degré se traduit pour la session 2022, par une baisse des rendements de concours d'environ 10% dans le 1er et le second degré. Le ministère a donc demandé aux académies. Lorsque des besoins apparaissent de mener une politique volontariste de recrutement de contractuels et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, pour effectivement pourvoir les postes vacants en leur proposant une rémunération cohérente avec celle des titulaires. Votre question elle renvoie plus généralement à la nécessaire. Attractivité et du travail sur l'attractivité du métier de l'enseignement des avec pour le ministère de l'Éducation nationale. Le chantier de l'amélioration de la rémunération des enseignants évoquée à de nombreuses reprises devant votre chambre d'autres métiers au sein du ministère sont également concernés. On pourrait être par exemple évoqué la revalorisation des militaires, des personnels de santé engagé depuis 2021 et qui se poursuivra en 2023. Mais globalement, l'amélioration des conditions d'exercice doit aussi permettre de renforcer l'attractivité et c'est donc tout l'objectif des concertations qui sont menées en ce moment par monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, monsieur Gilbert Roger. Vous voulez vous avez un peu de temps pour. je vais essayer de pas en prendre de trop. Merci, madame la Ministre. Je pense que il y a peut-être matière essayer de faire quelques évolutions parce que entre raté. L'Agreg à un point et ne pas avoir aucune proposition d'enquête dans la nature et organisée du speed dating comme ça a été fait dans l'académie des Yvelines. Pour trouver des gens qui n'ont aucune ambition première d'entrer dans l'éducation nationale. Je pense qu'il y a matière à pouvoir évolution donc s'il faut qu'on passe par la loi. Venant sera la loi mais je pense qu'il y a des évolutions que vous pouvez faire en votre qualité de ministre et d'adapter avec les recteurs, cela merci. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue. Cathy ah pour. Merci monsieur le président, madame la ministre, la colère gronde chez les enseignants, les parents, les élus la soustraction est devenue l'opération favorite du gouvernement pour le Pas-de-Calais. Ce sont 73 suppressions de classes et 53 suppressions de postes en primaire et maternelle, sans compter la la baisse drastique de la dotation horaire globale dans nos collèges et lycées qui induit la suppression de nombreuses options dans des bassins de vie durement touché par la crise sociale. De nombreux maires ruraux m'interpelle, qu'il soit d'ailleurs du bassin minier de la côte ou de la ruralité concernant la baisse des moyens dans l'éducation nationale qui entraîne de plus en plus de classes à triple niveaux voire quadruple parfois s'ajoute à cela le manque de remplaçants y y compris lorsque les absences sont prévues. Je suis surprise de la façon dont se déroule parfois le dialogue entre les maires et l'éducation nationale, pour ne prendre qu'un exemple récent, je citerai l'échange entre le RPI. le RPI. 2. Quénoi en Artois va Wakker yet et qu'hier un seul maire a été avisé du projet de fermeture de postes et pas le maire de la commune concernée d'ailleurs et lorsque les 3 maires du RPI ont écrit pour contester cette fermeture. Le rectorat leur répondez 10 jours plus tard que la décision a été validée sans avoir consulté la réponse des élus, les maires investissent beaucoup dans l'école, vous le savez quand quand car on ruralité. Il en va de la vie souvent du village de la même manière, faute de prise en compte des enfants de moins de 3 ans dans les moyens éducatifs à louer les écoles sont souvent dans l'incapacité d'accueillir les enfants en question. Les écoles sont le coeur de nos villes et nos villages, nous avons besoin de pérenniser l'école publique publique de proximité. Il est donc indispensable de fidéliser au plus tôt les familles cela suppose des moyens dédiés, et in fine et la prise en compte des moyens de moins des moins de 3 ans dans les tableaux d'effectifs je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Ah pour se. Dans le contexte que nous connaissons de forte baisse démographique tout dispositif. Visant à maintenir le service public de l'éducation partout dans le territoire est le bienvenu. À ce titre, les regroupements pédagogiques intercommunaux RPI demeure un outil d'aménagement scolaire très important à la rentrée 2022 4790 regroupement totalisant 9167 écoles sont recensées contre 4777 regroupement totalisant 9253 écoles à la rentrée 2021. En outre, 6997 communes sans école participe à un regroupement en légère augmentation par rapport à la, à la rentrée 2021 plus 66, regroupement soit près de 1%. Je me permets d'huîtres de saluer le travail des mères puisque pour pouvoir maintenir une offre scolaire sur le territoire, ils acceptent en lien avec les Dasen de former. De fermer certaines écoles et de former certains regroupements pour pour offrir des meilleures conditions d'enseignement aux élèves dans leur commune. Il convient de préciser que d'une manière générale, les travaux de préparation de la carte scolaire de rentrée donne lieu à de nombreux échanges avec les élus locaux et ont lieu sur la base d'une appréciation fine objective de la de la situation de chaque école et de ses de leur spécificité. Et de spécificité des territoires ce processus initié en janvier. Se poursuit jusqu'à la rentrée de septembre, dans un dialogue continu avec les élus et un suivi très attentif des évolutions éventuelles d'effectifs je termine en vous rappelant que les regroupements sont regardés avec une attention particulière compte tenu aussi des efforts de regroupement déjà réalisés par certains territoires. Je vous remercie. Merci la parole est maintenant à notre collègue Jean-Yves Roux. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Les écoles rurales accueil 36% des écoles métropolitaine et 20% des élèves. Elle répond à des 15. Tout à fait particulière, comme une forte propose sur deux classes multiniveaux soit 76% et des regroupements pédagogiques intercommunaux. Confronté à une Europe déprise démographique et à des difficultés de pérennisation des équipes pédagogiques, les élus ruraux mènent des politiques d'animations et d'attractivité pour que des familles et continue de faire la commune et leur pilier l'école. Or, chaque année, les élus sont confrontés aux coupures et de l'annonce des fermetures et ouvertures des classes fondée sur le seul critère des effectifs, la fameuse carte scolaire susceptibles de venir bouleverser des équilibres et dynamique locales conduite de haute lutte. Mes chers collègues. Les collectivités locales. Après l'état Après l'état les premiers financeurs de la dépense d'éducation. Malheureusement, le couple ne regarde pas ensemble dans la même direction en octobre 2019, mon collègue, le président l'a fort et moi-même avons présenté un rapport sénatorial portant sur les nouveaux territoires de l'éducation ce rapport soulignait que les écoles situées en milieu rural s'avère moins attractive pour les équipes éducatives et enseignante, c'est que ces élèves poursuivent des études dans des proportions bien inférieures à la moyenne nationale. Cela justifier une autre approche pour faire progresser la réussite scolaire. Parmi les propositions de ce rapport nous indiquant que le gel des cartes scolaires pendant 3 ans dans les territoires ruraux pouvaient apporter des réponses. Madame la Ministre, pendant ces 3 ans, les élus auraient eu le temps de mener des politiques publiques locales pour conforter leurs écoles et ses effectifs tandis que les équipes pédagogiques au réel aussi le temps d'installer des projets. Madame la ministre, il y a un an nous apporte d'options. La loi 3DS et qu'il entendait par la déconcentration rapprocher l'état du terrain, un soutien des collectivités. Nous sommes convaincus que l'éducation nationale gagnerait en efficacité, en s'inscrivant dans l'esprit de cette loi. Ma question, et c'est un peu madame la ministre. Allez-vous par expérimentation, tout d'abord proposer une carte ce Sollers stable valable pendant 3 ans pour la ruralité. Je remercie. Merci, madame la Ministre. l'engagement présidentiel de ne fermer aucune école de zone rurale sans l'accord préalable du maire de la commune a été pris. Vous le savez en 2019. Reconduit chaque année cet engagement concerne uniquement les écoles et non les classes et s'applique donc sans exception. Vous savez la démographie scolaire est en forte diminution. Malgré cette baisse qui est appelée à se prolonger, je tiens à le préciser, nous avons fait le choix de ne pas arrêter de ne pas nous arrêter à un simple travail arithmétique concernant la carte scolaire spécifiquement. En milieu rural où l'école publique constitue un élément de dynamisation du territoire. Ainsi, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte. Des différences de situation, notamment en matière économique territoriale et sociale à ce titre, elle est constituée d'indicateurs le respect des caractéristiques du réseau scolaire académique le maintien du service public dans des zones rurales et la réussite des élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées. Nous utilisons un indicateur territoriale qui intègre la typologie des territoires les des moins éloignés des zones urbaines au plus éloignés. Comme le préconisait votre rapport. D'autres dispositifs spécifiques sont mis en place en réalité je pense par exemple aux territoires éducatif ruraux que nous venons d'étendre à 10 académie compte tenu du volontarisme des élus locaux pour ce dispositif, mais je pense aussi à l'extension aux zones rurales de dispositifs d'accompagnement, telles que les cordées de la réussite. Qui maintenant qu'on ne près de 32.000 élèves dans dans les territoires ruraux, sur un total de 180.000 à l'échelle nationale ou encore l'école ouverte dans le cadre des vacances ah prenante. Depuis l'été 2020. Enfin, le dispositif des internats d'excellence. Est un levier important pour les élèves des territoires situés en zones rurales ou isolées. Je connais votre travail et votre engagement sur la question de l'organisation territoriale du service public de l'éducation, et soyez assuré monsieur le sénateur que nous continuerons à travailler en lien avec les élus locaux tous nos élèves à tous, à tous nos élèves d'accéder aux apprentissages dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Faisons attention aux collectivement. Deux minutes pour les réponses, parce qu'on a 44 question dans la matinée donc. La parole à notre collègue Antoine Lefèvre. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Le programme France travail jeune récemment appelé de vos voeux suscite doutes et inquiétudes parmi le réseau national des missions locales pour l'emploi. Ce projet qui se rattache au chantier France travail attendu pour 2024 prévoit de rebaptiser les missions locales sans pour autant leur maintenir l'exclusivité de l'accompagnement des publics accueillis les responsables des antennes locales voient ceci comme une volonté de l'État d'intégralement se substituer à eux sur le long terme, malgré leur forte implantation dans les territoires pour les publics en recherche d'emploi, engagé depuis plus de 40 ans pour l'insertion des jeunes, les missions locales se sont constamment réinventé. Pour suivre l'évolution des dispositifs d'insertion et fournir une offre sur mesure adapté au territoire et au public ciblé 6000 errements au dédoublement des objectifs entre les missions locales et Pôle emploi depuis le lancement du contrat d'engagement jeune en 2022. Cette annonce d'une double tutelle apparaît comme une menace pour le maintien des missions locales. Par ailleurs, les élus de l'Union nationale des missions locales avaient accueilli avec perplexité. L'annonce pour que l'attribution de l'opérateur, en charge du demandeur d'emploi se ferait désormais sur la base d'un algorithme conçu pour orienter sa recherche un moyen supplémentaire pour déboussoler encore davantage. Des publics précaires isolés pour certains et pour lesquels il convient de maintenir le lien essentiel de proximité avec le conseiller de missions locales. Ma question est simple, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser la portée véritable ce nouveau projet et nous apporter toutes les garanties sur la préservation de l'autonomie des missions et des moyens de nos missions locales. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre. il est proposé comme vous l'indiquez que les mises sur le, qui le souhaitent prennent la la la la l'appellation France travail jeune cela n'emporte évidemment pas qu'elle soit seule en charge de l'accompagnement vers l'insertion professionnelle de tous les jeunes. Les missions locales auront pour principal objectif de mettre en oeuvre les parcours d'accompagnement des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement global socio-professionnel, ce qui constitue un enjeu majeur pour l'insertion des jeunes, elles co-élaborent aux côtés de l'opérateur France travail. Une proposition de feuille de route pour l'ensemble du public jeune pour sur chaque territoire qui sera soumise à la gouvernance du comité France travail coprésidé par l'État et les collectivités locales à ce titre leur rôle et donc renforcer l'orientation sera réalisée sur la base de critères partagé. Qui permettront aux jeunes de bénéficier d'un diagnostic et d'un accompagnement pertinent ce qui conduira aussi à diminuer les effets de concurrence entre réseaux. Le contrat d'engagement jeune continuera d'être porté conjointement par les missions locales et pour l'emploi avec une orientation des publics en fonction des besoins des jeunes et dans le cadre d'un développement des complémentarités d'une coopération sur chaque territoire dans le cadre du ce contrat d'engagement jeune jeune en rupture, il s'agit également d'articuler les interventions des missions locales avec des structures retenues dans le cadre d'appels à projets le partage des offres de service. Le développement de commun numérique physique mais de la logique ou le soutien à la formation et au partage de pratique sur des territoires portés par le projet France travail contribueront à cette logique de coopération et de complémentarité. Par ailleurs l'État poursuit son accompagnement conséquent aux missions locales avec un montant de 600 millions d'euros. De crédits de paiement en 2023 et par ailleurs un financement et un soutien Adeline à l'UNM elle qui ont été renforcés de manière conséquence depuis 2022 pour organiser l'animation national des missions locales. Merci Monsieur Lefebvre vous voulez ajouter un mot. Oui, merci, madame la Ministre, pour ces précisions étant moi-même président depuis plus de 20 ans d'une mission locale qui a été fusionné à une maison de l'emploi de la formation je sais par expérience que les jeunes, les élus, les partenaires ont besoin de signaux clairs et d'une ligne de conduite simple et d'une prise en charge exclusive au plus près des territoires aujourd'hui encore près de 150.000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification. Ils ont besoin de nous et ce n'est pas un algorithme qui améliorera la prise en charge. Alors s'il vous plaît, faites confiance au réseau des missions locales. Merci. Merci je vais saluer Madame la Ministre Carole Granjean et accueillir. Madame la ministre Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. je pense que on va vous laisser vous installé près du micro. Et je vais tout de suite passer la parole à notre collègue Gilbert Luc devina. Merci monsieur le président. Madame la ministre ma question porte sur les contraintes juridiques qui restreignent. La mutualisation d'exploitations de la vidéoprotection entre plusieurs communes cette mutualisation présente de nombreux avantages comme l'augmentation des capacités d'investissement pour du matériel plus performant, la mutualisation des charges de personnel et le renforcement des territoires couverts par la vidéo pour la gouvernance d'une telle mutualisation peut être mise en oeuvre sous différents régimes comme la création d'un syndicat à usage unique ou une entente intercommunal par convention. Cette dernière solution offrent des avantages de souplesse sans augmenter le nombre de structures sur le un même territoire. Pour autant, elles sortent à des difficultés de mise en oeuvre qui réduit son attrait pour les communes intéressées. L'instruction gouvernementale du 4 mars 2022, laisse entendre que dans le cas d'une entente intercommunal l'exploitation des images des communes associées ne peut se faire que par un policier municipal si les communes décident d'affecter un agent technique communal ou un agent de surveillance de la voie publique. Ceux-ci ne pourraient à leur visualiser que les images de la commune qui leur énumère. Ainsi l'intérêt d'une telle multitude une mutualisation disparaît aussi serait-il possible dans une entente intercommunal de positionner en exploitation des opérateurs en vidéoprotection ou des agents de surveillance de la voie publique et non de réserver cela au sol policiers municipaux et d'ouvrir la possibilité à ses agents de visualiser les images du territoire de toutes les communes, membre de l'Entente intercommunale. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, devina. La loi sécurité globale préservant les libertés du 25 mai 2021 a apporté de nombreuses possibilités nouvelles pour développer la vidéo-protection et la mise en commun de police municipale. L'article 42 de cette loi a ainsi étendu la possibilité de visionnage d'images de la voie publique, issu de la vidéoprotection à des agents territoriaux qui ne relèvent pas des cadres d'emploi de la police municipale. Les agents communaux peuvent ainsi solliciter un agrément préfectoral afin de leur permettre de visionner les images de vidéoprotection de leur territoire communal. Si la loi n'a effectivement pas prévu de régime de mutualisation strictement pluri-communale de ses agents. Elle a autorisé la mise à disposition vers les communes d'opérateurs de vidéoprotection qui ne sont pas policiers municipaux par les EPCI à fiscalité propre compétent et par des syndicats mixtes dans les communes sont membres. Ces agents peuvent alors être habilitées à visionner les images d'un territoire regroupant plusieurs de ses communes membres. Il n'a effectivement pas été prévu que de communes mutualisent la vidéoprotection par simple convention en employant des opérateurs de vidéoprotection en lieu et place de policiers municipaux. Cette question n'a d'ailleurs pas été soulevée lors de l'élaboration de la loi, il semble nécessaire d'évaluer, d'abord l'efficacité de l'ensemble de ces nouveaux dispositifs à la main des communes pour assurer assurer leur vidéo-protection, avant d'envisager le développement d'un régime supplémentaire de mutualisation d'agents spécialement dédié à cette mission. Je vous remercie. Merci monsieur Davina. Il vous reste une quinzaine de secondes. j'entends votre réponse je la connaissais. Simplement on peut comprendre que des élus ne souhaite pas augmenter les structures sur leur territoire. On peut aussi comprendre que des élus ne souhaitent que les policiers municipaux soient plutôt sur le terrain et ils sont confrontés aujourd'hui à une difficulté de recrutement des policiers municipaux. D'où ma question d'ouvrir à des agents non policiers municipaux qui puisse surveiller, surveiller l'ensemble de la, de la vidéo des communes associées. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Laurent Burgat. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Une aire d'accueil des gens du voyage situé à Villeneuve les Avignon, dans le Gard rencontrent des difficultés avec certains usagers venus des pays de l'Est qui ici sédentarise et organise à divers trafics. Bien que j'en sois tenté l'objet de ma question n'est pas de traiter ici et maintenant les problèmes occasionnés car ces derniers des sites carrément des réponses circonstanciées et c'est là où le bât blesse. En effet pour aborder ces questions. Les élus ne savent plus vers qui se tourner, car certains d'accueil est géré par l'agglomération du Grand Avignon dans le département du Vaucluse. Oui, madame la Ministre, bien que gardoise. Les communes de Villeneuve-lès-Avignon et les Anglais sont membres de cette agglomération, située à la fois dans un autre département, mais aussi une autre région, la région sud. Donc ma question est la suivante, est très simple. Quel préfet ces communes dans l'hôtel à saisir pour régler ces problèmes-là, je voudrais remercier. Madame la Ministre. Si monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Burgos. Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi numéro 2000 tirer 614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. L'article 9 de cette loi permet aux maires, quelle que soit la nationalité des occupants de demander au préfet du département, de mettre en demeure les occupants et de quitter les lieux. Cette mise en demeure n'est possible que si le stationnement viole les dispositifs d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires cette occupation doit en outre porter atteinte à la sécurité et la tranquillité ou la salubrité publique en dehors de l'hypothèse du stationnement illicite le maintien de l'ordre public sur le territoire d'une commune relève en principe de la compétence du maire en tant qu'autorité titulaires du pouvoir de police générale toutefois en l'application de l'article L. 22 15 tirer 1 du code général des collectivités territoriales le préfet compétent pour prendre toutes mesures relatives au maintien de l'ordre public. Si aucune mesure n'a été prise par le maire, malgré une mise en demeure restée sans résultat. S'agissant de la commune de Villeneuve les Avignon comme vous venez de l'indiquer, elle est membre de la communauté d'agglomération du Grand Avignon cette communauté d'agglomération regroupe ainsi que le permet le code général des collectivités territoriales. Des communes appartenant à 2 départements différents. Son siège est situé dans le département du Vaucluse. Pour autant, c'est bien le préfet du Gard qui est compétent dans la mesure où la commune de Villeneuve les Avignon est situé dans le département du Gard. Je vous remercie.

pensais bien que c'était ma Madame. La préfète du Gard avec qui d'accès internationaux avec les élus qui était compétente mais par rapport à cette problématique là il y a un problème de sécurité mais il y a aussi notamment pour les aires d'accueil sont nus compétence à des agglo et la politique de la ville qui peut concerner est aussi une politique des agglo et c'est vrai que c'est très compliqué pour les nouveaux élus. D'arriver à trouver qui est compétent par rapport à ses compétences qui peuvent être des fois interférer sur divers départements et diverses régions mais je vous remercie d'avoir éclairé les élus des angles. Merci. Cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue François Bonhomme. Merci monsieur le président, madame la ministre je souhaite attirer votre attention sur la procédure de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Des communes qui subissent des phénomènes de retrait gonflement des argiles et sur le financement de la couverture de ce risque, vous le savez, ce phénomène touche près de la moitié du territoire national. Les conséquences sont souvent désastreux désastreuse timbre pour l'habitat individuel que pour les bâtiments publics qui connaissent alors d'importantes dégradations. Le coût de la réparation de sauvegarde des bâtiments s'avère très souvent impossibles à supporter pour les propriétaires singe une protection assurantielle lié à la reconnaissance de cet état de catastrophe naturelle. Un dédommagement est certes prévue par depuis 89 dans leur régime Catnat et la loi de 2000. Mais malgré cela la règle de mise en oeuvre par l'autorité administrative au point sur les demandes communales. Ça reste très insuffisante, seulement la moitié des communes concernées parviennent obtenir une telle reconnaissance. D'autre part, face à l'accroissement du phénomène RGA le fait le financement de ce risque. Hé bien évidemment posé son coût total est estimé à plus de 3 milliards d'euros dans les prochaines années. De plus, l'ordonnance du 8 février 2023 qui doit permettre d'augmenter le nombre de communes éligibles à cette reconnaissance limiterait les indemnisations aux sinistres les plus graves, ce qui ferait sortir certains propriétaires de la couverture assurantielle, dès lors, Madame la Ministre quelles dispositions complémentaires entendez-vous prendre afin que les communes concernées par le berger a puissent bien bénéficier de la reconnaissance de l'état de 400 naturel et que surtout, l'ensemble des propriétaires touchés soit éligibles à ne telle indemnisation des dommages sur le bâti, y compris lorsque certains d'entre eux décident d'abandonner. Leur habitation. Enfin dernière question, quel est le plan de financement envisagé pour maintenir. L'équilibre du régime Catnat. Pff. Merci. Madame la ministre. monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur bonhomme. L'indemnisation des dégâts provoqués par le phénomène de sécheresse réhydratation des sols est assurée par la garantie catastrophe naturelle. Conscient des limites des modalités actuelles de prise en charge des effets de ce phénomène. L'article 161 de la loi dite 3DS du 21 février 2022 a habilité le Gouvernement entreprendre par voie d'ordonnance. Une réforme des modalités d'indemnisation du phénomène sécheresse réhydratation des sols au sein du régime de la garantie catastrophe naturelle ainsi l'ordonnance 20 23 Du 8 février 2023 a prévu. Un assouplissement des critères pris en compte pour analyser le caractère anormal des épisodes de sécheresse. Deuxièmement, une prise en compte des communes ayant subi une succession anormal de sécheresse d'ampleur significative mais dans l'intensité mesurée, année après année n'est pas exceptionnel. Et troisièmement, une meilleure prise en compte la situation des communes adjacentes aux communes reconnues en état de catastrophe naturelle afin de répondre aux effets de bord des critères actuels. Elle prévoit également l'encadrement des modalités de réalisation des expertises diligentées par les assureurs qui sera assorti de contrôles et de sanctions pesant sur les experts des assureurs qui ne remplissent pas les exigences de qualité qui seront fixées par décret. Enfin, l'indemnisation sera concentrée sur les sinistres susceptibles d'affecter la solidité ou d'entraver l'utilisation normale du bâtiment endommagé. Le gouvernement souhaite accompagner en priorité les sinistrés, confrontés à des dommages matériels affectant la solidité de l'habitation ou susceptibles de générer des dommages graves à terme en outre l'ordonnance a prévu d'augmenter le nombre de communes éligibles à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Vous le voyez, le gouvernement est toujours pleinement mobilisés sur ce sujet, je vous remercie.

qui est prévu à à très moyen terme, je rappelle que le BRGM lui-même donc estime d'abord à 10 millions de d'habitation concernée. Et surtout que le il estime le coût cumulé de la sinistralité sécheresse à 43 milliards dans les 20 prochaines années, donc je veux dire, là on a vraiment on sera en mesure si on ne fait pas un effort de financement de réduire malheureusement encore plus le nombre de personnes qui puisse. Tomber sous ce régime de d'indemnisation. Merci cher collègue. La parole est maintenant à d'autres collègues Corinne Ferré pour la question suivante. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je souhaiterais vous interroger sur les délais de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports et des difficultés perdurant, dans le Calvados et plus largement sur l'ensemble du territoire national. Les Français ont davantage besoin de présenter un titre d'identité en cours de validité que par le passé. Or la crise sanitaire l'effet Brexit et l'augmentation structurelle de la demande ont pour conséquence un allongement des délais de délivrance. Actuellement, le délai moyen pour obtenir un rendez-vous en mairie serait de 58 jours hé bien plus dans certains territoires, particulièrement en zone urbaine. Malgré le plan d'urgence, lancé par le gouvernement en mai 2022, les résultats restent très insuffisants. Cette année ce sont près de 14 millions de Français qui doivent refaire leur pièce d'identité, soit 5 millions de plus que l'an dernier pour faire face à la, à la demande les collectivités vont certainement devoir embaucher, ce qui aura un coût de même forcé de constater que ce sont les élus locaux, les maires au 1er chef et les agents communaux qui sont les victimes collatérales des dysfonctionnements constatés confronté à la frustration des d'usagers agacé par les délais d'attente, il n'est pas rare qu'ils soient victimes de violences verbales, voire pire. Il semblerait qu'il y ait un véritable engouement également pour la nouvelle carte nationale d'identité sécurisée. L'été approchant les demandes vont aussi encore augmenter. Je souhaiterais donc savoir ce que le gouvernement entend mettre en oeuvre afin d'assurer un délai raisonnable de délivrance de titres de titres d'identité aux usagers. L'objectif de temps devant être aussi de garantir une offre de proximité pour tous sur l'ensemble du territoire national. Merci. Merci cher collègue. Madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Ferré en 2022 face à l'augmentation exceptionnelle des demandes de titres d'identité et concomitamment des délais en matière de délivrance. Le ministère de l'Intérieur des Outre-mer a mis en place de nouvelles mesures, l'accompagnement des mairies est une priorité, et les mesures prises doivent permettre de limiter les conséquences de l'augmentation continue de la demande sur leurs services. La définition de règles nationales de priorisation du traitement des demandes et de mesures dérogatoires favorable au passage d'examen avec un titre périmée depuis moins de 5 ans doit ainsi permettre de contenir le volume des demandes. Le moteur national de recherches de rendez-vous. Permet aux usagers de connaître les disponibilités sur une zone géographique donnée, et de réduire le nombre de rendez-vous non honorés. L'enregistrement d'une pré-demande en ligne est encouragé car il permet de limiter la durée des rendez-vous de recueil et d'augmenter le nombre de rendez vous assurer le soutien financier est également prévu grâce à la revalorisation exceptionnelle de la dotation Titres sécurisés pour porter l'enveloppe globale, à 73 millions en 2023 pour une plus grande proximité avec les usagers. 500 nouveaux dispositifs supplémentaires sont en cours de déploiement et seront déployés à fin avril. Cette nouvelle augmentation significative de communes pouvant accueillir les demandes des usagers va contribuer à la réduction des tensions que vous relevez La récente loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer prévoit d'affecter des effectifs supplémentaires pérennes. Le suivi attentif du maillage territorial en. Et l'accompagnement donc dispositifs traduit l'engagement du gouvernement à garantir un service de proximité de qualité pour tous les usagers sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Merci madame un Ministre de votre réponse. J'ai été alertée par plusieurs maires de mon département, le Calvados, qui m'ont fait part de leur inquiétude, voire des difficultés qu'il rencontre depuis plusieurs mois. Alors les nouveaux moyens que vous annoncez nécessiteront aussi un peu de temps, du temps d'installation des machines, du temps de formation des agents. Il y a urgence car nos concitoyens sont en attente depuis trop longtemps maintenant, merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Pierre Vogel. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre promue par le gouvernement. L'habitat inclusif défini par la loi Elan de 2018 fait l'objet d'un financement particulier la prestation d'aide à la vie partagée. Il est destiné aux personnes handicapées ou âgées qui choisissent un mode d'habitation individuelle qui garantissent inclusion sociale à vie autonome tout en restant au domicile la demande et on peut le comprendre croissante et le regroupement de plusieurs personnes handicapées est indispensable pour la mutualisation des prestations financées par le conseil départemental l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe a développé depuis 1994 un habitat inclusif de 16 logements adaptés aux personnes handicapées moteur aux caractéristiques PMR plus plus dont chacune bénéficie d'un bail d'habitation à titre personnel dans un immeuble de 25 appartements au total. Or la commission de sécurité du SDIS de la Sarthe a requalifié l'immeuble en établissements recevant du public. Se fondant sur un arrêté de 1980, au terme duquel la présence de plus de six personnes en situation de handicap, dans un même immeuble emporte de facto cette qualification. Le bailleur social propriétaire n'ayant pas réalisé les travaux d'adaptation de l'immeuble dans les délais impartis. Le maire du Mans a prononcé la fermeture administrative et tous les occupants se trouvent menacés d'une expulsion imminente, aucune solution de relogement adaptée n'en trouver pour les occupants handicapé. Il y a donc incompatibilité entre les réglementations ERP et habitat inclusif regroupant plus de 6 logements pour PMR avait des conséquences lourdes probables classification ne RP de tous les habitat inclusif nouvelles fermetures administratives menace d'expulsion. Coup d'arrêt à l'habitat inclusif Madame la Ministre quelles dispositions urgentes entend prendre le gouvernement pour sauvegarder l'habitat inclusif existants, ainsi que permettent son développement. Envisagez-vous de soutenir financièrement les bailleurs publics et privés afin qu'il prévoit la création de logements adaptés à l'habitat inclusif six maximum. Sans doute pour échapper à la qualification de RP dans toute construction nouvelle afin de permettre la mutualisation des prestations handicap et d'imposer peut être aussi un certain nombre de logements destinés à l'habitat inclusif pour chaque chaque nouvelle construction. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Vogel, le cadre général de la sécurité incendie des locaux d'hébergement relèvent de la réglementation relative aux habitations porté par le ministère en charge de la construction. Cependant la réglementation relative aux établissements recevant du public ERP relevant du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer peut s'y substituer afin de garantir la sécurité des usagers. Dès lors qu'ils sont à l'extérieur de leur domicile internat scolaire hôtel et cetera ou que l'aptitude de ceux-ci ne leur permettrait pas de se soustraire seul aux effets d'un incendie l'habitat inclusif, qui est une solution de logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Alternative à l'habitat individuel, isolé et à la vie collective en résidence fait actuellement l'objet d'échanges interministériels visant à concilier la préservation du lien social avec l'impérieuse nécessité de protéger nos populations les plus fragiles et particulièrement exposés lors d'un incendie. Dans le cas cité en exemple le bâtiment concerné comporte 15 logements répartis dans des étages accueillant des personnes infirmes moteurs cérébraux reconnues comme des personnes handicapées sévère les privant d'autonomie pour accompagner les actes de la vie quotidienne en application de la réglementation, la sous-commission départementale de sécurité a proposé au maire après une visite sur place en avril 2022 le classement en ERP, le propriétaire n'ayant pas mis son bâtiment en conformité avec la réglementation. Le maire a pris un arrêté de fermeture le 8 décembre 2022 qui a fait l'objet d'un contentieux administratif, le Conseil d'État a confirmé par une ordonnance du 20 février 2023, le statut de RP de ce bâtiment, en s'appuyant notamment sur la situation de fragilité des résidents, les porteurs de projet doivent donc intégrer que l'autonomie du public accueilli, est un des critères déterminants du statut juridique de l'établissement. Je vous remercie. Merci la parole est maintenant à notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne. Merci beaucoup monsieur le le président, madame la ministre ma question porte sur la situation des communes limitrophes ou proches des zones de revitalisation rurale ces zones de revitalisation rurale cette enfin c'est un dispositif qui est indispensable pour un certain nombre de collectivités, près de 18.000 d'entre elles en France sont concernées avec des avantages fiscaux sociaux pour conforter leur attractivité. Pour autant, il y a un certain nombre de communes qui sont situées à proximité et qui. Est bien du coup, rencontre des difficultés pour attirer un certain nombre de professionnels, je pense à des professionnels de santé parce que c'est vrai que le régime. Intéressant. Dans les communes ZRR voisine fait que ces professionnels peuvent être tentés dévisser leur plaque et donc. Ma question est simple, a été de savoir quels étaient les les dispositifs les réflexions qui était en, en cours au sein du gouvernement pour peut être. Trouver. Comment dire amoindrir l'effet frontière l'effet seuil. Et faire en sorte que ces communes. Qui rencontrent aussi des besoins. Et d'attirer des professionnels ne soit pas desservie par la présence voilà d'une zone. Plus attractive à côté. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Lemoine. Les zones de revitalisation rurale, les ZRR sont dispositif d'exonération fiscale et sociale, vous l'avez dit visant à favoriser l'attractivité des territoires ruraux. Parmi ces aides un dispositif d'exonération fiscale pour les médecins généralistes exerçant dans une commune en ZRR est effectivement présents comme vous l'indiquez, et comme c'est le cas pour la plupart des dispositifs de zonage des effets frontière peuvent exister. Le dispositif ZRR prend fin au 31 décembre 2023, depuis l'été 2022. Je travaille sur l'avenir des ZRR ce travail repose sur une mission que j'ai confiée au préfet François Philizot, avec le soutien de la direction générale des collectivités locales, la DGCL les effets de bord de frontières inhérents aux ZRR sont bien identifiés, notamment en matière de déserts médicaux et un des objets de cette mission et d'y apporter une solution. Cette problématique rejoint aussi pour partie, celle des communes rurales qui ne sont pas classées en ZRR car appartenant un EPCI n'étant lui-même pas classées en ZRR. Nous travaillons donc un mécanisme permettant par dérogation à l'application d'une méthode national de calcul au niveau des EPCI de faire entrer certaines communes dans le dispositif dès lors qu'elles émargent aux critères de zonage. Ainsi, dans les semaines qui viennent. Des annonces seront faites sur l'avenir des ZRR à partir de janvier 2024 mais également sur une nouvelle déclinaison de l'agenda rural sous l'appellation générale de France ruralité ces annonces trouveront leur place dans un plan national ambitieux à destination des territoires ruraux, plan qui tiendra bien évidemment compte des problématiques que vous évoquez en y apportant des solutions concrètes et adaptées aux problématiques de chaque territoire. J'aurais à leur plaisir à vous le présenter, je vous remercie.

Je sais que les collègues ici Delcros espagnol qui ont également travaillé permettra de conforter ce régime et que vous pourrez effectivement trouver des des modalités pour les communes riveraines voisines. C'est exactement le sens. Des déclarations qui avait fait en son temps le préjudice Jean Castex lorsqu'il s'était déplacé Migennes dans l'Yonne et qu'il avait été sensibilisés par monsieur le maire. À cette époque et le Premier Ministre s'était. Montré ouvert à travailler à des dispositions qui pourraient trouver leur place en prélève ou PLFSS et donc voilà. Nul doute qu'avec les orientations que vous avez évoquées. Nous allons continuer le travail et je l'espère aboutir. Merci. La parole à notre collègue Bruno Belin. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je voudrais qu'on revienne quelques instants sur la loi notre. La loi note ça ça a été un, un véritable séisme pour un certain nombre de collectivités. Je pense aux départements qui ont perdu la clause de compétence générale qui ont perdu la compétence économique qui ont perdu une des compétences de proximité les plus symboliques était le transport scolaire qui ont été transférés à à des grandes régions qui évidemment n'essaie avait moins la connaissance du terrain, grande région sur lequel il y aurait beaucoup à dire puisque déjà le constat qui est fait depuis 7 ou 8 ans, c'est qu'aucune économie de fonctionnement n'a été fait avec ces grandes régions qui ont gardé parfois leur hôtel de département de de régions dans dans d'anciennes capitales régionales et ça a été un, un vrai séisme mais ça a été un cataclysme. Pour les collectivités locales, et sans doute les collectivités locales les plus rurales, parce qu'on les a fait rentrer parfois contre leur gré. Dans des. Établissements publics de coopération. Communal de grande taille communautés urbaines. Moi j'ai plusieurs exemples dans la Vienne autour de Poitiers ou mécaniquement. Évidemment leur potentiel financer a doublé, triplé alors que évidemment les maires s'interrogent et se dise. Ma population est pas venu de plus riche. Conséquence immédiate, effondrement. De la DGF et vous avez aujourd'hui des communes qui sont asphyxiés dans l'élaboration de leur budget qui sont en train d'essayer de leur faire qui ne sont pas capables. J'ai des exemples en tête de pouvoir mener un budget d'investissement parce que leur budget de fonctionnement et le boucle pas et donc je pense à ces communes aujourd'hui comme lignée

Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Belin. Le potentiel fiscal et le potentiel financier communales ont pour vocation de retranscrire de la manière la plus objective possible en neutralisant les choix budgétaires et de gestion des collectivités locales. Le niveau de ressources Libre d'emploi qu'une commune est en mesure de retirer à la fois de la fiscalité locale et de la fiscalité transférée qu'peut percevoir mais aussi la richesse qu'elle tire de son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre PCI. En effet, au sein d'un EPCI, il a fait ce qu'elle était propre, une commune bénéficie directement ou indirectement, des produits de fiscalité économique des prélèvements. Fiscaux intercommunaux ou bien encore de la répartition des attributions de compensation décidée par le conseil communautaire ce mode de calcul commun à l'ensemble des communes appartenant à un EPCI faisant application du régime de la fiscalité professionnelle unique, ce qui est le cas de 90% des communes assure la comparabilité comparabilité de leur niveau de ressources potentielles entre elle et constitue la condition sine qua non d'une répartition objectif et équitable des différentes composantes de la DGF au niveau national. Je vous rejoins cependant sur le fait que le niveau local joue un rôle essentiel pour assurer une plus grande solidarité entre les communes. Il dispose pour cela d'outils dédiés plusieurs mécanismes fiscaux permettent en effet d'assurer une plus forte péréquation des ressources vers les communes les moins dotées, telle la révision Libre des attributions de compensation ou l'institution d'une DSC dotation de solidarité communautaire. J'ajouterais également qu'il existe un dispositif de répartition locale de la DGF dont les élus peuvent se saisir afin de définir des règles de réallocation des attributions DGF qui leurs sont notifiées avec l'ensemble de ces outils, les collectivités ont donc la possibilité de faire jouer la solidarité intercommunale, je complète en disant que je suis à votre entière disposition pour poursuivre ces échanges. Je vous remercie.

Le pic ce fonds de péréquation. Il faut l'unanimité du Conseil que communautaire. Donc, c'est chaque fois ça ne marche pas, donc il faut absolument trouver les moyens de créer des fonds de compensation pour sauver les communes rurales. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant. À notre collègue Cédric Vial. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre. Ma question concerne le dispositif du zéro articulations nettes, disant inscrit dans la loi de 2021. Dites climat résilience lequel impacte directement les collectivités territoriales, dans son discours de clôture du congrès des maires. Madame, la Première ministre a confirmé l'objectif de 2050 pour la des artificialisation des sols. Elle a également précisé que les objectifs devaient être territorialisées et différenciés, sans trahir les ambitions nationales. Elle a également indiqué que les projets d'envergure nationaux seront décomptés à l'échelle nationale. Ces annonces sont des éléments importants pour les collectivités toutefois des questions subsistent par exemple en Isère. L'entreprise STMicroelectronics ça a annoncé une extension de son usine qui permettra de doubler la capacité de production avec à la clé la création de plus de 1000 emplois sur place. Ce projet rentre dans la stratégie de la politique nationale de soutien de la filière électronique et en terme de développement industriel comme le président de la République a pu le préciser. Lui-même lors de son déplacement sur le site de cette entreprise. Toutefois, pouvez-vous nous dire si cette extension sera décompté à l'échelle nationale et quel décompte sera prise en compte uniquement le tellement foncier de cette extension ou aussi les conséquences de l'arrivée 2000 nouveaux salariés sur le territoire. En effet, ces créations d'emplois vont se traduire par des logements supplémentaires des services publics équipements complémentaires seront-ils intégrés dans le décompte si ce projet n'est pas pris en compte au niveau national ces conséquences impacterait a minima l'enveloppe foncière disponible de 3 Scott différents ce qui empêchera quasiment toute autre forme de développement endogène. Or, une augmentation de leur enveloppe ne pourrait être envisagée qu'en révisant à la baisse la capacité de développement des autres Scott régionaux pour conserver les les objectifs à l'échelle du sera Fradette qui devra lui aussi être modifié compte tenu des délais de mise à jour de ses multiples documents, l'entreprise devra attendre plusieurs années avant de pouvoir déposer un permis de construire, alors. La réactivité nécessaire pour notre autonomie industrielle si nos entreprises doivent attendre l'évolution de ces documents Khadr pour déposer. Un début de projet sera mise en cause l'intervention des différents documents sera dette Scott et PLU pourrait même rendre tout projet important de ce type impossible à être mise en oeuvre. Merci, cher collègue, la parole à Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Vial. Vous avez interrogé. Monsieur Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et ne pouvant être présent il m'a chargé de vous répondre. La Première ministre a réaffirmé l'objectif national d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'Hénaff d'Hénaff sur la décennie 2021 2030, la préservation des sols est en effet nécessaire pour stocker du carbone et préserver la biodiversité nous protéger face aux impacts du changement climatique. Vous évoquez plus spécifiquement la problématique des grands projets nationaux. Le gouvernement s'est à plusieurs reprises exprimé sur le fait qu'il souhaitait que les projets d'envergure nationale ne soit pas décompté à l'échelle de chaque région. Mais à l'échelle nationale afin de permettre une mutualisation des efforts. Cette mesure est en cours de discussion dans le quart de la proposition de loi sénatoriale sur Lausanne concernant les projets économiques jugés d'intérêt national. Une réflexion est en cours sur leur périmètre avec des évolutions possibles dans le cadre du projet de loi industrie vers porté par mes collègues Bruno Lemaire et Roland Lescure. Par ailleurs, la loi climat et résilience organise déjà la possibilité d'avoir recours à une mutualisation au niveau régional des projets d'envergure. Vous proposez que soit identifié les besoins induits par les projets d'ampleur nationale aux régionales en terme d'infrastructures, d'équipements ou de logements connexe au projet lui-même disproportionné conduirait à prendre en compte des projets qui peuvent relever exclusivement d'enjeux et de considérations locales sans présenter d'enjeux régionaux supra. Régionaux le Sénat n'y est pas favorable, les amendements que vous avez porté sur le sujet. N'ayant pas été adopté. Je vous remercie. Merci madame la ministre et la parole est maintenant à notre collègue Olivier Cigolotti. Merci monsieur le président. Madame la ministre ma question concerne le dispositif MaPrimeRénov qui rencontrent actuellement de nombreux et importants dysfonctionnements. Cette mesure gouvernementale encourageant la rénovation énergétique. Des logements et l'éradication des passoires thermiques à inciter les ménages et les entreprises, le plus souvent artisanales à se lancer dans des travaux importants. Cette incitation financière a généré une forte augmentation du nombre de dossiers cependant du fait des difficultés rencontrées par l'Agence nationale pour l'habitat, l'Anah opérateur en charge de la gestion et la logistique de la distribution de ces primes. Les entreprises, tout comme les particuliers sont souvent toujours en attente du versement des montants alloués par MaPrimeRénov. Cette situation leur est extrêmement préjudiciable et ses bénéficiaires sont contraints d'effectuer des avances répétées de trésorerie qui deviennent très dur à supporter. Certains se trouvent même confronté à des négociations difficiles avec les banques pour soutenir leur trésorerie et dans les cas les plus extrêmes à la perspective d'une cessation d'activité. Au vu de la situation, il ne s'agit pas d'incriminer telle ou telle structure mais simplement d'alerter sur une situation qui devient de plus en plus préoccupante dans un certain nombre de départements dont le mien, la Haute-Loire, les difficultés de versement de MaPrimeRénov remettent en cause l'existence même de certaines entreprises et pénalise également les ménages, notamment les plus modestes. quelles mesures le gouvernement entend mettre en oeuvre afin d'accélérer et de sécuriser le versement de cette prime indispensable à l'accélération de la rénovation énergétique du parc de logements français Merci madame la ministre, à vous la parole. MaPrimeRénov en matière de rénovation énergétique et la principale aide de l'État pour accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique. Cette dernière a permis de soutenir plus de 1,4 millions d'usagers. Depuis son lancement en janvier 2020. Dans un contexte de forte demande et de montée en puissance du dispositif certaines demandes ont pu rencontrer des difficultés et aboutir dans les délais habituels. Excusez-moi. Dans un contexte de forte demande et de montée en puissance du dispositif certaines demandes. Puis rencontrer des difficultés à aboutir. Dans les délais habituels. Toutefois, le nombre de cas est très limité l'se mobilise très fortement pour fluidifier le parcours usagers avec la mise en place d'une équipe dédiée aux situations les plus difficiles. Les dossiers en difficulté font l'objet d'un suivi individualisé pour résoudre au plus vite ces situations-là n'a, mais tous les moyens nécessaires en oeuvre pour assurer la qualité et la rapidité du traitement des dossiers. Le délai moyen de traitement pour un dossier MaPrimeRénov est inférieur à cinq semaines pour un dossier complet et ne nécessitant aucun contrôle renforcé. Il est environ de deux semaines. Pour une demande de subvention et d'environ 3 semaines pour obtenir le paiement lorsqu'un dossier nécessite des documents justificatifs complémentaires ou fait l'objet d'un contrôle sur place pour lutter contre la fraude. Ces délais peuvent être allongée et peuvent atteindre 3 mois. Il ne s'agit donc pas de nier les difficultés. Mais de leur ramener à juste proportion dans un dispositif dans le succès est indéniable et qui est un pilier de notre politique de rénovation énergétique. L'amélioration de l'information aux usagers est également une priorité avec l'objectif d'accompagner l'augmentation du volume de projets de rénovation. La création du service public France rénove en 2022, complété par la montée en charge progressive de mon accompagnateur rénove en 2023 permettra de faciliter le parcours des ménages dans leur projet de rénovation. Je vous remercie. merci Madame la Ministre pour votre réponse. Mais ce dispositif MaPrimeRénov a suscité beaucoup d'intérêt par les possibilités qu'il offrait en termes de de travaux de rénovation énergétique. Mais il est aujourd'hui, source de grande déception tant à cause des délais de paiement que des difficultés opérationnelles qu'il génère. vous en avez convenu, il est plus qu'urgent de de fluidifier le le traitement de ces dossiers en attente et et pour les dossiers à venir je vous remercie. Merci la parole est maintenant à notre collègue Vincent second. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je reviens vers vous au sujet de la suppression des moulins et des seuils et notamment le cas précis d'décès de l'Orne, dont certains sont aujourd'hui fortement menacé par les arrêtés pris en préfecture. Même si le gouvernement a prétendu vouloir s'engager pour la sauvegarde de notre Patrimoine. Il apparaît néanmoins qu'il reste des domaines dans lesquels les actes ne sont pas à la hauteur des attentes relatives à la préservation des monuments historiques et culturels de nos territoires. Ce manque de considération à l'égard de notre héritage le conduit tout droit sa stricte disparition pire que cela. Cette absence de politique de préservation, gens de la destruction volontaire de bon nombre de monuments historiques qui font la fierté l'honneur et l'histoire de nos territoires. Cette situation s'est particulièrement illustré dans mon département de l'Orne, avec la commande de le l'effacement du seuil de la bataille d'exercice sur l'Orne en 2010 par le préfet et ce sans discussion cet effacement a eu lieu, alors même qu'il avait été proposé au préfet de la direction départementale des territoires. Un projet de micro centrales hydroélectriques par la réhabilitation d'un bâtiment historique dont l'origine remonte au XIIIe siècle. Ne nous en sommes pas remis de nombreux me Moulin faisant encore partie de secrétaire Gauri est en passe d'être détruits. Je m'interroge logiquement aujourd'hui sur la constance de l'engagement du ministère à ce sujet ou sur le respect de la parole ministérielle dans les administrations de nos départements alors que ces dernières n'ont pas suivi la réponse à leurs formulée par vos prédécesseurs lors des 2 précédentes questions que j'en avais déjà adressé à ce sujet le gouvernement m'avait pourtant assuré de la sauvegarde des moulins à forte valeur patrimoniale aux producteurs de petite hydroélectricité. 3 questions Madame la Ministre, pouvez-vous me dire quelle orientation suivez-vous en terme de continuité écologique de préservation du Patrimoine et de production propre. Si ces politiques sont bien partagées par l'ensemble des ministres qui sont concernés et enfin l'information est-elle relayée auprès des préfets des administrations compétentes, merci. Merci, madame la Ministre. Avec la politique de continuité écologique en effet le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, travaille avec le ministère de la culture pour identifier les ouvrages sur lesquels une thématique patrimonial nécessite une attention particulière des effacements ou écrasement de Moulins. On peut avoir lieu dans l'ordre et dans d'autres départements, sans que cela soit contradictoire avec la sauvegarde du Patrimoine. Ces opérations ne touche en général qu'au seuil Dumoulin et peuvent être l'occasion de rénover des éléments clés du Moulin concernant le seuil de la bataille de clefs si la solution mise en oeuvre a fait l'objet d'une concertation au sein de la commission locale de l'eau du sage Orne moyenne conformément aux recommandations de ce sage la auteur de l'ouvrage a été réduite en ce qui concerne la production d'électricité des moulins. Les débats sur la loi d'accélération des énergies renouvelables a rappelé ont rappelé que leur contribution était modeste dans le mix énergétique et qu'elle ne peut justifier les atteintes aux milieux aquatiques pour finir depuis août 2021, la loi interdit aux services de l'État de prescrire l'effacement d'un moulin en réponse à l'obligation de rétablissement de la continuité écologique des consignes en ce sens ont bien été passé et sont respectées néanmoins un propriétaire peut toujours demander l'abrogation de son droit d'utiliser la force motrice de l'eau et souhaité la remise en état du cours d'eau plutôt que d'aménager continuer à supporter les charges d'entretien d'un seuil en rivière qui peut être coûteux et chronophage. Il n'appartient pas au service du ministère de s'opposer à une telle requête de la part du propriétaire exerçant son droit je vous remercie. Je vous ai bien entendu un ministre seulement ce ne sont pas les propriétaires qui sont en demande d'arasement des des seuils ce sont ce sont les. les organismes de sauvegarde. De la continuité écologique qui demandent les rarement de ces de ces seuils, peu importe la valeur patrimoniale ou peu importe l'hydroélectricité. Ce que vous venez de dire. Parce qu'on considère que c'est pas assez un traumatisme auprès des populations et des propriétaires qui est majeur et on voudrait juste avoir une administration qui soient compréhensifs qui écoute et qui soit objective. Et qui soit une

Haropa première 1er port commercial de France. En fait la route stratégique de notre politique exportatrices françaises relais entre la capitale et la façade maritime française l'axe Seine est aussi un outil majeur pour la réindustrialisation française. Cela s'illustrent par son inscription en 2019 dans territoires d'industrie qui accueille aujourd'hui plus de 20% de l'ploie industriel en France. Mais que ce soit dans les boucles ou dans son estuaire. La scène est concernée elle aussi par le principe de zéro artificialisation nette l'application stricte Dusan en Seine Maritime illustrent bien les contraintes majeures qui seront imposées à nos territoires face aux besoins fonciers importants

bloqueront demain toute initiative de l'axe Seine car inclus dans le compte foncier des territoires sur lesquels ils sont implantés. Sans compte foncier séparés pour l'axe Seine. La ligne nouvelle Paris-Normandie ou les projets, développement. Logistique d'repas seront à l'arrêt, tout comme Port-Jérôme. À Port-Jérôme sur scène les problèmes rencontrés sont aussi ceux de la compensation environnementale et ou de l'absence de volet fiscal incitatif à la réutilisation des friches. Alors ma question est simple, Madame la Ministre comptez-vous clairement inscrire dans la loi les comptes foncier dans les dans les comptes foncier nationaux les opérations d'aménagement dans les circonscriptions portuaires. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Chaque année, 20.000 hectares d'espaces naturels agricoles et forestiers. 20.000 hectares sont consommés en moyenne en France, les conséquences de ce phénomène sont écologiques, mais aussi socio-économiques. En effet, la France s'est fixé l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation des Naf dans les 10 prochaines années. La loi climat et résilience organise déjà la possibilité pour la région de mutualiser à son niveau des projets d'envergure comme ceux portés par Aarau. La Première ministre s'est déclaré favorable à une évolution législative, de sorte que les projets d'envergure nationale ne soit pas décompté à l'échelle de chaque région mais bien mutualisés. À l'échelle nationale de cette manière les territoires concernés ne seront pas pénalisés par leur implantation. Le gouvernement a présenté dans le cas de l'examen de la proposition de loi sénatoriale un amendement visant à intégrer explicitement les grands ports dans les grands projets d'envergure nationale. La rédaction intègre ainsi dans ses projets. Les actions ou opération d'aménagement réalisés sur leur territoire par un grand ports maritimes ou fluviaux maritimes de l'État ou pour leur compte. L'objectif de sobriété foncière est ambitieux mais nécessaire pour accompagner les territoires à s'engager en faveur de la sobriété foncière plusieurs aides sont déjà déployés, que ce soit à travers le renforcement de l'ingénierie territoriale l'encouragement à la contractualisation où la mobilisation de leviers fiscaux ou budgétaires, en particulier le Fonds Vert qui a été dotée en 2023 de 2 milliards d'euros. Je vous remercie. Merci madame. Une quinzaine de secondes. Oui merci Madame le Ministre ne nous trompons pas, il y a pas de remise en cause de l'enjeu de sobriété foncière. On est bien d'accord mais il ne faut pas décourager. Les les utilisateurs par l'inscription dans leurs comptes foncier de Denges d'envergure nationaux

Madame la ministre, à la ligne ferroviaire de l'Aubrac est une ligne emblématique du Massif central, elle relie Clermont-Ferrand à Béziers et dessert les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Lozère, de l'Aveyron de l'Hérault. Et cette ligne joue aussi un rôle essentiel pour le tissu économique en assurant le fret pour l'usine ArcelorMittal situé à Saint-Chély-d Apcher qui est le 1er pourvoyeur d'emplois du secteur sa portée symbolique et son intérêt touristique sont également très fort puisqu'elle franchit le célèbre viaduc de Garabit construit par Eiffel qui fait l'objet d'une demande de classement au Patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'elle traverse les gorges de la hier actuellement classé et faisant l'objet d'une opération grand site de France. Autant d'atouts qui ont conduit l'État à renouveler classement cette ligne en train d'équilibre du territoire jusqu'en 2031, reconnaissant ainsi son intérêt national. Malgré les travaux réalisés pour sauvegarder cette ligne l'absence d'anticipation et d'entretien sur certains tronçons ont conduit à sa fermeture durant 11 mois en 2021 Et, selon plusieurs sources, la ligne pourrait à nouveau fermer dans les mois à venir si des travaux n'était pas engagé rapidement notamment sur le tronçon situé dans le Cantal, en train de la et Baresse, alors Madame la Ministre face à cette incertitude, nous avons besoin d'être rassurés sur la cohérence des politiques de l'État classé une ligne ferroviaire d'intérêt national et la fermer faute d'entretien ne serait ni cohérent ni acceptable aussi. Pouvez-vous nous assurer que la ligne de l'Aubrac ne subira pas de nouvelle fermeture par défaut d'entretien ou de travaux non effectués. Et du coup, pourriez-vous nous indiquer le calendrier des travaux envisagés pour l'éviter. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Delcros. L'État est pleinement engagée aux côtés des régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes en faveur des deux lignes interrégionales de l'Aubrac et des Cévennes auquel sont associés de forts enjeux financiers territoriaux pour les territoires qu'elle traverse, l'État a ainsi intégralement tenus les engagements financiers qu'il avait pris sur ses 2 lignes au titre des CPER 2015 2022 afin de maintenir leurs performances. L'État a par ailleurs fait des propositions aux deux régions pour assurer le financement dans la durée des lourds investissements nécessaires à leur sauvegarde dans le cadre d'un projet de protocole d'accord inter-régional destiné à donner une visibilité à 10 ans et à définir une stratégie de long terme pour ces 2 lignes. Je suis à ce jour en attente de leur réponse. À plus court terme sur la ligne de l'Aubrac, le remplacement de certains rails de type le double champignons entre Neussargues et Saint Chély la psyché doit être effectuée rapidement afin de pérenniser les circulations ferroviaires de voyageurs et de fret sur cette section, je vous confirme que l'État est prêt à mettre en place sa part de financement pour réaliser cette opération. Des discussions sont encore en cours entre les deux régions Oxygen Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour compléter le tour de table financier de ces travaux prévus en 2024. Je vous remercie. Madame la Ministre. D'une façon plus générale le réseau des petites lignes ferroviaires ne doit pas être regardée comme relevant du passé. Elles sont une chance pour notre pays et peuvent nous aider à répondre à des enjeux majeurs, la lutte contre le réchauffement climatique. Cette ligne est entièrement électrifiés surtout son parcours mais aussi répondre à des questions de mobilité en milieu rural et je sais que vous y êtes sensible. Donc s'il vous plaît, ne laissait pas tomber ni cette ligne de l'Aubrac, ni les petites lignes, le Massif. D'ailleurs à la chance de disposer d'un réseau assez intense assez dense plutôt Michel de petites lignes ferroviaires. Merci. Et maintenant, la parole est à notre. Martine Filleul. Merci monsieur le président, madame la ministre ma question porte sur l'aéroport de Lille-Léquin si sa modernisation est nécessaire son extension, fait l'objet de vide vive inquiétude et de rejet de la part des habitants et des élus des communes avoisinantes. L'ARS a alerté sur l'effet des nuisances sonores que produirait l'augmentation des vols de nuit sur l'apprentissage scolaire les troubles du sommeil et les risques d'infarctus. Face à ces menaces sur la santé, la qualité de vie des 550.000 des 55.000 riverains, comme le préconise l'ARS. Il est absolument nécessaire d'instaurer un couvre-feu la nuit, de 23h à 5h du matin. C'est une mesure de bon sens et de responsabilité qui s'applique déjà aux autres aéroports Beauvais hors ligne Nantes ou encore Bâle Mulhouse, alors pourquoi pas aussi à Lille un cela fait plusieurs mois que le gouvernement est saisi de cette question par les parlementaires, par les élus mais aussi par la population à chaque occasion vous l'esquiver. En prenant l'engagement de la mise en place d'une mesure d'impact d'une étude d'impact, mais elle n'est même pas nécessaire pour prendre la bonne décision préconisée par tous les experts, à savoir la mise en place d'un couvre-feu. Alors je vous pose très directement la question Madame la Ministre allez-vous oui ou non instaurer un couvre-feu visant à protéger et garantir la santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice filleul. L'objectif affiché par le syndicat mixte, propriétaire de l'aéroport de l'île Léquin le s'Malim et par son exploitant et de porter le trafic de passagers de l'aéroport de de 2 millions en 2019 à 3, 4 millions en 2039. L'ambition initiale qui était de 3,9 millions a été réduite compte tenu des changements de pratiques des passagers utilisant l'avion en raison de la restructuration de la compagnie Hop à la sortie de la crise sanitaire qui a conduit au maintien d'une seule ligne régulière vers Lyon et à l'abandon des dessertes de Bordeaux, Nantes, Marseille, Nice et Toulouse. Le trafic s'est élevé à 1,8 millions de passagers en 2022, pour un nombre de mouvements commerciaux de 13.683, mouvement contre plus de 20.000 en 2019. Concernant les vols de nuit le s'Malim et l'exploitant ont pris l'engagement de plafonner le nombre de vols de nuit à celui de 2019, soit 1566 mouvement or les vols d'avions et de de l'État et les vols sanitaires, une étude d'impact, selon la méthodologie de l'approche équilibrée a de plus été lancée à la demande du ministre chargé des Transports sous le pilotage du préfet du Nord imposée par la réglementation nationale avant la mise en place de toute mesure de restrictions d'exploitation sur un aéroport comme celui de Lille comprend des analyses socio-économiques et des étapes de concertation de l'ensemble des parties prenantes du territoire. Elle permettra de déterminer les mesures de réduction du bruit et d'éventuelles restrictions d'exploitation adapté à la situation locale et proportionnée. D'un point de vue socio-économique dans ce cadre une large concertation sera organisée avec un point d'avancement prévue lors de la réunion de la commission consultative de l'environnement qui aura lieu en juin prochain. Je vous remercie. Merci. Une quinzaine de secondes Madame. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre vous me faites un début de réponse qui ne correspond pas du tout à ce que j'attendais sur la dimension économique de la modernisation. Je vous l'ai dit, elle est la bienvenue. Cette modernisation. Mais pour ce qui concerne le plafonnement des vols de nuit. La réponse n'est pas satisfaisante quant à l'étude d'impact, mais écoutez j'accepte l'augure d'une étude d'impact mis en place en juin mais sachez que les populations aussi bien que les élus du territoire sont très impatients de l'avoir mis en place. Merci cher collègue. Et je passe maintenant la parole à notre collègue Jean-Raymond Hugonet. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre de l'association drapeau présidée par Monsieur Gérard Bouthier et qui défend les riverains de la plateforme aéroportuaire d'Orly rassemble à ce jour plus de 30 communes et 30 associations riveraines de l'aéroport. À leurs côtés nous militons depuis plus de 20 ans pour une exploitation rationnelle de celui-ci. Cette approche vise à prendre en compte la protection de la santé, le respect des droits des populations survolées ainsi que les impératifs d'une activité territoriale responsable et durable. Le 12 juillet 2021. Nous avons appelé à l'application du règlement européen qui établit les normes et procédures pour la réduction du bruit des grands aéroports ce règlement exige que les États désigne une ou plusieurs autorités compétentes indépendantes de toute organisation participant à l'exploitation de l'aéroport. Or en désignant la direction générale de l'aviation civile comme autorités compétentes l'État français ne se conforme pas à cette règle d'indépendance. Aussi, dans son arrêté, rendu le 5 avril 2022, le Conseil d'État a reconnu que la DGAC n'était pas impartial et a demandé à la Première ministre de nommer une nouvelle autorité indépendante dans les 6 mois. Pourtant voilà 10 mois que la DGAC et toujours juge et partie. Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer pour quelle raison l'injonction du Conseil d'État n'est-elle pas suivi d'effet. Merci cher collègue Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Hugonnet vous appelez notre attention sur la pollution sonore engendrée par le trafic de l'aéroport de Paris Orly le trafic sur l'aéroport de Paris Orly et d'ores et déjà soumis à un ensemble de contraintes à visée environnementale qui font l'objet d'une surveillance stricte par les auto rité local de l'aviation civile depuis 1968 un couvre-feu est en vigueur entre 23h 30 et 6h du matin, l'aéroport fait l'objet d'un plafonnement à 250.000 créneaux par an. Le plan de prévention du bruit dans l'environnement ppb propre à l'aéroport qui a été adoptée le 17 mars 2022 et par ailleurs, le seul plan qui prévoit un objectif de réduction du bruit. Quantifier. Il s'agit de diminuer d'au moins 6 décibels, l'indicateur moyenner de gêne sonore ressenti en période nocturne entre 22h et 6h et réduire de 50% le nombre de personnes affectées par de fortes perturbations du sommeil parmi la population exposée au bruit aérien sur la même période. Une étude d'impact, selon l'approche équilibrée en application du règlement, UE. 598 2014. Étudiera les mesures et restrictions d'exploitation complémentaires qui pourraient être mises en place pour atteindre cet objectif. Comme vous le soulignez. Le Conseil d'État a par une décision du 5 avril 2022 remis en cause le rôle de la direction générale de l'aviation civile, en tant qu'autorités compétentes en matière d'étude d'impact, selon l'approche équilibrée. Un projet de décret portant désignation d'une nouvelle autorité compétente est actuellement soumis à l'examen du Conseil, l'aboutissement de cette réforme est un préalable indispensable. À la réalisation de l'étude d'impact que j'évoquais, je vous assure que le gouvernement est attaché aux politiques publiques liées à la lutte contre les nuisances sonores. Je vous remercie. termes galants ces choses là sont dites madame la ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous. L'État français bafoue une décision du Conseil d'État. Nous avons 6 mois et vous avez six mois madame, la Première ministre pour désigner quelqu'un, ce n'est toujours pas le cas. C'est cela que nous attendons. Et la réponse que vous nous donnez éteint. Encore une fois, excusez-moi, sans attaques personnelles mettant un sabir technologique. Ce que nous attendons, c'est la décision ferme et définitive d'une autorité totalement indépendante, ce qui n'est pas le cas de la DGAC. Merci de analyse. Merci. Donc nous allons continuer. Et la parole est maintenant à Pascal à la présidente. Pascale Gruny, je crois que c'est Madame la Ministre qui va continuer à répondre aux questions. Si j'ai bien compris.

vais je vais suspendre quelques secondes hein. On va reprendre tout de suite le temps.

la séance et et reprise et donc je, je donne la parole pour sa question à la présidente. Pascale Gruny. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre un article du Parisien daté du 8 février 2023 évoquent un désaccord entre les médecins et la Haute Autorité de Santé concernant l'efficacité de certains traitements ciblés contre le cancer. Ces traitements dispose d'une autorisation de mise sur le marché et selon les médecins, ils ont fait leurs preuves dans le cadre d'essais cliniques. Cependant, la Haute Autorité de Santé estime que les données cliniques dont elle dispose aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour considérer que le service médical rendu justifie une prise en charge par la solidarité nationale face à la maladie, tous nos concitoyens doivent pouvoir bénéficier des meilleurs traitements. Il en va de leur confiance dans notre système de santé et de sécurité sociale. Dès lors, pourquoi la Haute Autorité de Santé considère tels que ces traitements de devrait pas être remboursé par la Sécurité sociale, nous avons besoin de comprendre ces décisions pour mieux les accepter. Madame la ministre de la Haute Autorité de santé dispose-t-elle aujourd'hui réellement des outils nécessaires pour appréhender ces nouvelles thérapeutiques. Merci, madame la Ministre, que je remercie de répondre à la question. les éléments suivants, en réponse à votre question. L'évaluation des produits de santé en France et en Europe vise à garantir que les médicaments autorisés sur le marché présente un niveau d'efficacité suffisant et un profil bénéfice-risque. Jugé favorable au vu des alternatives disponibles afin que les patients. Puisse en retirer un bénéfice. La prise en charge des produits de santé, en particulier des médicaments repose en France sur une double exigence d'une part identifié parmi les médicaments de profil bénéfice-risque jugé favorable les médicaments présentant un niveau d'efficacité justifiant leur prise en charge et identifié dans le cadre d'accès précoce. Les médicaments pour lesquels la présomption de bénéfices et suffisamment forte pour justifier une prise en charge. D'autre part permettre à l'ensemble des patients éligibles. L'accès à ces médicaments. La HAS. Est chargé de manière collégiale et en toute indépendance d'évaluer pour chaque médicament demandant son remboursement par l'assurance maladie, son service médical rendu l'amélioration du service médical rendu. Qu'il apporte par rapport aux alternatives exigeante. Son niveau d'exigence est élevé, en particulier concernant les données soumises par les industriels en vue de cette évaluation des études cliniques comparatives randomisée en double aveugle reste ainsi un prérequis néanmoins il peut exister des situations particulières dans lesquelles ces études sont impossibles. La Commission de la transparence a fait évoluer ses modalités d'évaluation pour tenir compte de ces situations particulières. En ce qui concerne les traitements pour lesquels la HSS. H A S a conclu à une absence de cela ne s'assimilent pas à un refus de remboursement puisque ces traitements s'ils sont à destination du secteur hospitalier sont pris en charge au travers des tarifs hospitaliers enfin certains traitements font l'objet d'autorisation de mise sur le marché disent dites conditionnel ce qui signifie que le rapport bénéfice-risque n'a pas encore été confirmée de manière certaine et que l'Agence européenne du médicament conditionne cette autorisation à la collecte de nouvelles données pour confirmer cette présomption de bénéfice Par ailleurs, il faut souligner que notre système national de prise en charge précoce des médicaments. Permet un accès aux traitements présumés innocents innovants pour les patients souffrant de maladies graves et rares pour lesquelles il n'y a pas d'autre traitement approprié disponible en France ce système unique permet aux patients français d'accéder aux traitements les plus innovants, avant même qu'il ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Même la ministre. Là ce sont des médecins. Qui ont réagi, donc des médecins qui expérimentent eux aussi les les mes médicaments dans on les essais cliniques, donc on ne parle pas seulement des patients là en fait il révèle une perte de chance et surtout on je crois que nous sommes dans l'Union européenne si ces médicaments sont homologués en Europe et pas en France et quand on voit aussi le sujet aujourd'hui de la pénurie de médicaments qui est quand même en partie liée aussi au prix bien entendu ces médicaments innovants sont plus chers. Donc on peut se poser la question quand même si il y a pas cette question financière et je trouve que quand on parle de santé, ce n'est juste pas possible. La perte de chance et inexplicable pour les patients, donc j'espère que le ministre entendra cette cette question et cette demande qui n'est pas à à tourner d'un revers de main. Merci. Merci madame la présidente. Donc nous remercions la Ministre Dominique Faure et nous accueillons. Madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé pour les questions suivantes. Et je passe tout de suite la parole à notre collègue François Bonneau. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Le Conseil économique, social et environnemental a entamé la la publication des résultats du vote organisé à la suite de la 2ème phase de la convention sur la fin de vie. En février 2023. 75% des personnes et citoyens interrogé se sont prononcés en faveur d'une aide active à mourir. Qu'il s'agisse du suicide assisté ou l'euthanasie. Aux personnes majeures ou mineures, sans que le pronostic vital ne soit nécessairement engagée. Toutefois la la loi 2016 87 du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ainsi qu'un rapport du comité consultatif d'éthique, publié en 2022, suggère que l'aide à mourir doit être circonscrite à des conditions strictes telles qu'une affection grave et incurable ou bien lorsque le pronostic vital est engagé. Ces conditions sont également l'objet de nombreuses législations étrangères. Dont on parle régulièrement ou l'aide à mourir, a été encadré, Belgique, États-Unis, Autriche, Pays-Bas. Même si l'accompagnement de la fin de vie doit faire l'objet de réformes, au vu du mal mourir la mauvaise prise en charge de la souffrance mettent également en lumière des inégalités d'accès aux soins palliatifs. Selon un rapport du Sénat, publié en 2021, 26 départements ne disposait pas d'unités de soins palliatifs. Ou d'au moins un lit pour 100.000 habitants en 2019 aussi, j'aimerais connaître la position du gouvernement sur la fin de vie et le droit à mourir et plus spécialement à la question porte sur quelle politique seront mises en oeuvre pour améliorer l'accompagnement de la souffrance en fin de vie, notamment pour renforcer l'accès aux soins palliatifs. Merci cher collègue là, madame la Ministre. Merci monsieur le président, monsieur sénateur, vous le savez, le président de la République a souhaité que nous ayons collectivement un débat sur la fin de vie. Des travaux sont engagés à différents niveaux par la Convention citoyenne par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat par la Cour des comptes et enfin par le gouvernement, moi-même en lien avec Olivier Véran. Nous avons ainsi à proposer à des parlementaires de chaque groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat mais aussi à des professionnels de santé reconnu de participer à nos travaux dans le cadre de débats thématiques sur l'anticipation et la culture palliative mais aussi l'accompagnement du deuil et la reconnaissance du rôle des aidants en fin de vie. Ces travaux constituent le terreau d'une future stratégie d'accompagnement de la fin de vie que j'appelle de mes voeux concernant l'accès aux soins palliatifs il apparaît d'ores et déjà nécessaire d'envisager une feuille de route pour renforcer notre politique en terme de développement des soins palliatifs et d'accompagnement à la fin de vie. J'ai demandé en ce sens à ce que la procédure de rénovation de la circulaire de 2008 relative à l'offre de soins palliatifs déjà ancienne et pour partie obsolète soit engagé sans attendre en outre une 3ème édition de l'Atlas des soins palliatifs vient d'être publié, il souligne les progrès réalisés en terme d'installation d'unités de soins palliatifs. Si 20 départements ne dispose pas aujourd'hui l'unité de soins palliatifs, cela ne ne signifie pas pas pour autant qu'il n'y a pas d'offre de soins palliatifs sur ces mêmes territoires les cartes présentées par département souligne en effet, le nombre d'équipes mobiles de 100 palliatifs dont 171 sont déployés sur l'ensemble du territoire national, de lits de soins palliatifs en établissement sanitaire comme en services de soins de suite et de réadaptation. Au fil des auditions que j'ai pu mener de mes déplacements dans les territoires aller et à l'étranger dans les services de soins palliatifs comme au domicile de certains malades et des dents. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des soignants des personnels des bénévoles très investi ému par une profonde humanité. Si beaucoup a été fait. Je souhaite qu'un nouveau cap soit passée pour assurer une intégration active effectif à même de répondre aux besoins des Français. Vous l'aurez compris, le dialogue national sur la fin de vie est loin d'être achevée. Mais quel qu'on soit l'issue, il faut garder à l'esprit le caractère profondément singulier douloureux et complexe de chaque situation. En fin de vie. Je vous remercie.

Je ne doute pas de de de votre volonté mais vous savez que dans les pays où la législation est la plus avancée. Les unités de soins palliatifs ont été parfois et les grands perdants de ces situations donc c'est pour ça que je vous le. Cette attention toute particulière pour une situation que vous avez évoqué, qui est effectivement à la fois très douloureuse et très particulière. Merci. Cher collègue, la parole à notre collègue Laurence Arribagé. Merci monsieur le président, madame la ministre ma question porte sur l'impact du prix des médicaments sur la situation des entreprises productrices de médicaments mature en France. qui sont doublement pénalisés actuellement par l'inflation. Et qui augmente les coûts des intrants et de l'énergie couplée à une réglementation toujours plus contraignantes sur les prix des médicaments et puis sur la pression des prix fixés par un accord cadre avec le comité économique des produits de santé. Or chaque année les Budgets couvrant l'achat de ces médicaments matures sont revus à la baisse. De fait, la situation financière de ces entreprises et de plus en plus précaire. Or notre souveraineté sanitaire et l'accès des médicaments à nos concitoyens dépendent beaucoup de de de ces entreprises. Comment cette la disposition qui demande au c'est au PS de de de fixer le prix en prenant en compte l'impératif de sécurité d'approvisionnement est effectivement mis en oeuvre aujourd'hui. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Le Ministre de François Braun regrette de ne pouvoir être présent ce matin la tarification d'un médicament s'appuient majoritairement sur sa valeur clinique notamment son niveau d'amélioration du service médical rendu dit à SMR, un nouveau critère de tarification a été créé par la FSS 2022 pour mieux prendre en considération la sécurité d'approvisionnement du marché français qui garantit l'ampli dans l'implantation industrielle afin d'appliquer concrètement ce nouveau critère le CE PS. Élaborer une doctrine de critères d'éligibilité et de niveau de valorisation récemment finalisé cette doctrine peut dorénavant être mise en pratique pour les entreprises commercialisant des produits essentiels lorsque niveau de prix ne serait plus compatible avec la garantie d'un maintien sur le marché. L'article 28 de l'accord-cadre signé entre le PS et les industriels permet d'accéder à une hausse de prix. Si les critères d'éligibilité prédéfini sont réunis. Les postes de surcoût considéré sont aujourd'hui ceux liés à la matière première toutefois un élargissement de ce périmètre au surcoût lié à la production dans sa globalité, pourraient être considéré, pour des médicaments de fortes criticité sanitaire et industriels. Une liste de médicaments stratégiques d'intérêt sanitaire et par ailleurs en cours d'élaboration avec les sociétés savantes afin de définir les molécules pour lesquelles le levier du prix pour être actionnée. S'il s'avère pertinent pour assurer leur maintien sur le marché. Finalement, une mission interministérielle sur les mécanismes de régulation et de financement des produits de santé a été lancée sous l'égide de la Première ministre en janvier dernier, dont les conclusions sont attendues pour l'été prochain 2 des principaux objectifs annoncés dans le cadre de cette mission sont le renforcement de notre tissu productif, notamment pour les produits matures essentiel dans un objectif de souveraineté sanitaire l'attractivité des territoires pour les industriels et la relocalisation de produits de santé stratégique. Ainsi, le gouvernement est pleinement mobilisée autour de l'enjeu prioritaire qui est la manière de réguler le prix du médicament pour faire face aux enjeux actuels de demain.

parce que l'article 28 ne prévoit une hausse du prix des que lorsque l'arrêt de la production de la commercialisation empêcherait de couvrir un besoin thérapeutique, comme vous l'avez dit alors qu'il s'agit ici de garantir la diversification des approvisionnements, lors d'une récente audition avec Pascale Gruny mon interlocuteur me confiait que qu'une seule augmentation de prix avaient été consentis pour un montant de 2 centimes la boîte. Il ne faut pas oublier que le CE PS et placée sous la tutelle du gouvernement et donc il est de votre responsabilité et j'espère que cette mission dont vous avez fait. Référence permettra d'aller beaucoup plus loin parce que la question est vraiment très importante. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Guy Bénard Roche. Merci monsieur le président, madame la la ministre dans le cas de la stratégie d'investissement Ségur de la santé des priorités ont été ciblés sur mon département des Bouches-du-Rhône. Cette volonté de réinvestir dans notre système de santé est une réelle opportunité pour notre territoire avec une occasion de moderniser nos infrastructures d'adapter ses capacités, ses services à l'évolution démographique à l'horizon 2030 de 1050. Hé bien au-delà ce doit être également l'occasion d'anticiper sur les métiers et les personnels qui seront nécessaires. Cependant, depuis sa mise en oeuvre et les différents projets du Ségur font face à une forte inflation de leur coup avec une augmentation des prix, notamment de l'énergie et des matières premières. Les hôpitaux concernés ne peuvent pas co-, financer les projets prévus puisque tous lourdement déficitaire vivant déjà sous la perfusion financière des aides de l'ARS. Si, a-t-il d'exemple dans les Bouches-du-Rhône les de construction de centres hospitaliers de Salon-de-Provence avec un apport de 78 millions de l'ARS pour un projet estimé à 130 millions et Aubagne avec un apport de 92 millions de la RS pour un projet estimé à 115 millions font face matelas des surcoûts de 30% environ ses projets devient difficilement soutenable et il est demandé par exemple pour le projet d'Aubagne qui initialement devait être encore plus de la santé de revoir à la baisse ses orientations par exemple en retirant la partie médico-social du projet et aurait étudiants surdimensionnement actuellement le projet est estimé à 140 millions d'euros, sans le médico-social. Nous devons de répondre. Aux besoins de santé des habitants vivant dans les communes concernées. À proximité, y compris dans celles du Var proche d'Aubagne grâce à centre hospitalier moderne au service au nombre de lits adaptés aux besoins et facilement accessible. C'est une réelle de mode de tous les maires de ce territoire. Nous ne pouvons pas construire un nouvel hôpital uniquement au regard du budget mais davantage en fonction des besoins en santé de la population pour les 50 prochaines années à venir. Je vous demande donc de préciser le montant du soutien financier supplémentaire de l'État sur ses projets à la suite de ces surcoûts et de garantir que les besoins de santé des habitants de ces territoires notamment à moyen et long terme seront bien pris en considération pour déterminer l'apport financier de l'État. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Cette situation appelle une certaine prudence de la part des porteurs de projets et l'obligation pour eux de reconsidérer l'estimation de leurs opérations pour tenir compte de ces nouveaux coûts de construction et provisionner des aléas économiques cohérent avec l'inflation prévisionnelle les réévaluations s'élève effectivement pour les projets que vous citez à environ 30% par rapport aux données de la programmation initiale au Ségur investissement. Le ministère de la Santé est conscient que les établissements peuvent difficilement absorber cette augmentation des coûts ainsi des alternatives sont en cours d'analyses pour identifier des sources de financements complémentaires qui permettraient d'équilibrer leur plan de financement des collectivités locales ont ainsi pu être sollicité de nouveau dans les ARS. Des travaux sont menés sur le rééchelonnement possible de certains projets. S'agissant plus particulièrement de celui d'Aubagne. Il s'agit du projet de reconstruction pour lequel l'aide provisionnels de l'ARS est le plus élevé en région PACA. En effet le CH Edmond Garcin occupe une place importante dans l'offre sanitaire de proximité de l'Est des Bouches Rhône que nous entendons consolider la situation financière dégradée de l'établissement a conduit l'ARS a positionné un niveau d'accompagnement prévisionnel très important dont le montant sera définitivement fermé au moment de la validation du projet. Ainsi, afin de prendre en contres ces évolutions, le projet médical et le projet immobilier sont actuellement en cours de consolidation et de lieu à de nombreux échanges avec l'établissement en lien également avec les services de la préfecture et de la direction départementale des territoires de la mer. C'est dans ce contexte que le choix a été fait de privilégier une approche différenciée entre un volet sanitaire et un volet médico-social de ce projet en particulier ce qui pourra entraîner un décalage dans le calendrier des 2 volets afin de poursuivre la réflexion autour de l'organisation future de l'offre médico-social local en lien avec les autres acteurs du territoire cette réflexion intègre la question de l'implantation des sites de la recomposition de l'offre et du développement d'une offre innovante. Il ne s'agit pas dont il ne s'agit donc pas d'aéroport si dédié du volet médico-social mais d'une maturation de la réflexion afin de prendre en compte les spécificités propres au développement d'un tel projet qui dans la configuration actuelle de la situation nécessite d'avoir lieu séparément dans un calendrier dédié tout en permettant aux projets sanitaires de progresser pour répondre aux besoins de la santé. Merci madame la ministre. La parole est maintenant à notre collègue Ronan Le Gleut pour la prochaine question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre la réforme dite Puma instaurant la protection universelle maladie a des conséquences particulièrement néfastes pour les Français établis hors de France. Récemment, j'ai été saisi de la situation d'une personne en situation de handicap. Dans l'incapacité de travailler, une française qui réside en Argentine avec ses parents retraités dont elle était l'ayant droit majeurs. Elle vient d'être brusquement désaffiliés, de la sécurité sociale et se trouve sans la moindre couverture sociale si des soins lui sont nécessaires. Lors d'un séjour en France. Cette situation touche également de nombreuses femmes qui n'ont que peu ou pas travaillé ayant suivi leur mari ayant accompagné leur carrière à l'étranger. Elle se retrouve notamment à l'heure de la retraite, elles aussi confrontées à la même difficulté. En effet, avant la réforme le statut d'ayants droit majeurs permettait aux personnes qui ne remplissait pas les conditions, notamment les épouses ou les personnes en situation de handicap, sans activité professionnelle d'être affiliés à l'assurance maladie généralement par le biais de leur conjoint ou d'un des parents eux-mêmes affiliés à la sécurité sociale. La réforme Puma a supprimé ce statut. Or, la suppression de ce statut a créé une situation profondément injuste pour nos compatriotes résidant hors de l'Union européenne dans les pays sans convention bilatérale de sécurité sociale ou ceux et où la convention bilatérale n'inclut pas pas les membres de la famille ainsi bouleversant subitement un modus operandi de plusieurs décennies. Cette réforme a pour conséquence que les anciens ayant droit qui réside dans ces pays ne peuvent plus bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé lors de leur court séjour en France, sauf à prendre une assurance supplémentaire auprès de la CFE-, la caisse des Français de l'étranger, ce qui double quasiment le montant de leurs cotisations. Cette loi donc des effets pervers et non anticipés pour les Français établis hors de France. Je souhaiterais savoir quelles mesures le gouvernement compte prendre pour que nos compatriotes qui réside dans ces pays continuent à bénéficier de la protection de l'assurance maladie lors de leur séjour en France. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre. pour justifier de la stabilité de sa résidence en France une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle doit fournir un justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Certaines catégories de personnes n'ont pas à justifier de cette condition. C'est le cas notamment des membres de familles qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France en assurer d'un régime de Sécurité sociale obligatoire français. L'article 206 tiré de du code de la Sécurité sociale établi une liste des catégories de personnes qui peuvent accéder à la prise en charge des frais de santé, sans répondre aux critères de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois. Bien que les Français de l'étranger ne soit pas mentionnée en tant que telle dans cet article, ils peuvent dans certaines conditions bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé dès le retour en France. Enfin, il convient de rappeler que la Puma n'a rien modifié le critère de résidence stable Dispositif qui précédait à la Puma prévoyait déjà la condition à la résidence stable en France depuis plus de 3 mois. La mise en place de la Puma a au contraire introduit une simplification des démarches de l'assuré et des ayants droit pour mieux garantir la continuité des droits de l'assuré en terme de prise en charge de ses frais de santé. de santé. La ministre, la parole est désormais à notre collègue Jean-Baptiste Leblanc. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre à Carpentras dans le Vaucluse, l'hôpital ou plutôt la partie service public du pôle santé public-privé. Va devoir fermer la nuit. Compte tenu de l'application de la loi Rist le 3 avril prochain et peut-être même définitivement. De de ses unités, les urgences et la maternité, l'intensification ces dernières années du recours à l'intérim médical ont conduit à une surenchère en matière de rémunération. Outre l'impact financier majeur dans les Budgets des établissements. Il s'avère que les plannings de garde sont aujourd'hui très dépendant de ses médecins. Ils représentent 40% des praticiens à Carpentras. Ces derniers ne souhaitant pas poursuivent leur mission au tarifs imposés, soit 1170 euros brut par mission de 24h et préférant se diriger vers les établissements privés, les hôpitaux se retrouvent à 15 jours de l'application de la loi Rist dans une situation insoluble. Faire un planning était déjà un casse-tête le faire en avril sans intérimaire et une mission impossible pour les chefs de service, tous les services, service d'accueil des urgences et SMUR gynéco obstétrique anesthésie-réanimation pédiatrie médecine sont désorganisés. À ce jour les habitants du compte avait naissance, c'est-à-dire 90.000 personnes hors saison touristique 200.000 en été sont systématiquement dirigés vers l'établissement centre d'Avignon, qui est déjà submergée. Aujourd'hui c'est qu'arpentera qui arpentera qui fortement impacté mais qu'en sera-t-il demain à Cavaillon Apt orange ou Vaison-la-Romaine. L'ARS se dit pleinement mobilisée pour éviter ce scénario catastrophe, mais quelles sont réellement ses moyens pour agir. Demain, l'heure n'est plus aux discussions autour de la revalorisation des salaires des praticiens hospitaliers qui aurait dû être fait il y a bien longtemps, l'heure n'est plus à discuter autour du numerus clausus, il faut trouver des médecins et ce avant le 3 avril. Aujourd'hui c'est toute l'offre de soins dans le Vaucluse où ces hôpitaux de proximité joue un rôle primordial qui est désorganisé par la mise en oeuvre de la loi Rist la proximité constitue pourtant un enjeu majeur d'efficacité de la médecine d'urgence avec la connaissance du terrain et des acteurs concernés, gage de chances pour les patients, madame la Ministre, les praticiens hospitaliers, les infirmiers, les pompiers, les médecins les Carpentras tient tout simplement hé bien au-delà des Vauclusiens attendent des garanties de l'État le 3 avril au soir, chaque mot aura-t-il encore accès un service d'urgence en moins de 30 minutes, je vous remercie. Merci madame la ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur. Vous évoquez les dispositions relatives à la régulation de l'intérim. Concernant l'application de la loi du 26 avril 2020, dite loi Rist assurer à chacun de nos concitoyens des soins adaptés et accessibles localement constitue une priorité pour le ministère de la Santé. Notre politique n'est pas de lutter contre l'intérim qui peut parfois représenter une solution à certaines situations de tension conjoncturelle en ressources humaines mais contre ces dérives qui mettent en péril l'équilibre de notre système de santé. C'est un poids financier majeur pour l'hôpital public avec certaines rémunérations pouvant atteindre 6000 euros pour 24h, cet argent c'est celui des Français. Nous n'acceptons pas qu'il puisse servir à entretenir ce type de dérives, c'est autant de moyens en moins pour revaloriser les carrières hospitalières, ces situations engendrent une profonde iniquité vis-à-vis des praticiens qui s'investissent durablement à l'hôpital. La loi prévoit déjà depuis 2016 un plafonnement des rémunérations à 1170 euros brut par 24h. Cette loi n'est pas appliquée et les infractions n'ont cessé de se développer. La loi Rist prévoit la mise en place de contrôles pour la faire respecter plusieurs fois répéter reporter l'échéance retenue pour la mise en place et le 3 avril 2023. Il est de la responsabilité du ministère de la santé que de faire appliquer la loi votée par le représentant de la nation et d'oeuvrer à la reconstitution des collectifs de travail dans les hôpitaux. Face aux difficultés transitoires que nous avons anticipé les ARS travaillent avec le réseau des finances publiques et les établissements pour mobiliser tous les acteurs publics comme privés afin de maintenir la continuité des soins. Des solutions alternatives au cas par cas sont travailler dans chaque territoire en fonction du contexte local dans une logique de solidarité territoriale, les collectivités territoriales et élus locaux sont des maillons essentiels de la réussite des politiques de santé. Une organisation dédiée à un thé a ainsi été mis en place au sein du ministère pour identifier les situations particulièrement signalé par les élus, nous étudierons en lien avec les ARS et leurs délégations territoriales toutes les situations de blocage qui nécessitent une attention ou une intervention particulière pour Carpentras. Depuis plusieurs années le CH fait appel à des vacations médicales pour compléter le tableau de garde et assurer la continuité des activités d'urgences de maternité mais également de médecine, la mise en oeuvre de la loi Rist constitue un changement important qui nécessite de revoir les rémunérations des médecins vacataires le CH met régulièrement en oeuvre des plans de continuité des activités lors de certaines périodes de tension, notamment durant les congés d'été de fin d'année des leviers RH vont être mobilisés par autorisation du DG augmentation de la prime de solidarité territoriale recours à l'emploi contractuel au titre de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre pour les territoires et enfin des adaptations organisationnelles seront nécessaires. Merci, madame la Ministre, même si je vous rappelle que le, le principe c'est deux minutes pour la la réponse. Bon. Donc faites attention parce qu'on a, on a encore beaucoup de questions dans la matinée. Merci. La parole est notre notre collègue Stéphane Le Rudulier. Merci monsieur le le président Madame la Ministre le le dialogue entre l'exécutif et les élus locaux sont toujours aussi compliqué, je le regrette profondément. Le couple mère préfet vantée par le président de la République en novembre dernier dans le cadre du salon des des maires apparaît dans les faits. Peu inopérant. La fermeture de nature plus ou moins arbitraire et sans aucune concertation des élus locaux de l'Epad intercommunal de la Durance situé dans les Bouches-du-Rhône et plus précisément sur le site de cabane en et, si besoin est une nouvelle illustration. Je ne suis pas ici pour contester le fond de la décision mais bien la forme, c'est-à-dire le manque de considération des élus locaux mais également du personnel de santé et surtout des pensionnaires dans cette prise de décision. En effet, le maire de la commune a appris cette fermeture le 16 novembre dernier par communication orale orale du directeur depuis ce jour, force est de constater qu'aucune communication officielle de la, de la part de l'ARS n'a confirmé la dite fermeture néanmoins, aujourd'hui, nous sommes devant le le fait accompli puisque la totalité des résidents du site de la maison de retraite ont d'ores et déjà été transférés sur un autre site d'accueil et au-delà du choc psychologique pour ces résidents. La commune de cabane, propriétaire du bâti dorénavant inoccupé a la lourde responsabilité de proposer un projet de réaffectation de cette structure sans accompagnement de l'État et sans une quelconque indemnité de compensation, faute d'avoir été impliqué dans la décision. De surcroît, la commune est frappée de plein fouet depuis plusieurs années par la désertification des services publics et après avoir perdu son bureau de poste en 2020 cette décision unilatérale s'apparente aujourd'hui à une double peine pour cette pour une petite commune de 4400 habitants alors Madame à Münich. Confirmez-vous de manière officielle, la fermeture du site de cabane de l'Epad intercommunal et si oui, êtes-vous en mesure de proposer un plan d'accompagnement et de soutien aux élus locaux. Quant à la future destination de ces bâtiments. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur, la situation de la maison de retraite publique intercommunal des communes de cabanes et nos Weiss hé bien connu des équipes du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées qui la suivent depuis de nombreux mois. Je sais à ce titre-que des échanges ont cours régulièrement au niveau local avec l'ARS le directeur général de la direction départementale des Bouches-du-Rhône avait ainsi adressé en date du 19 janvier 2023, un courrier à monsieur Gilles Mourgue, maire de cabane, difficultés, les difficultés de l'établissement n'était ni récente ni conjoncturelle et ouvrant sur une proposition de rencontre déjà concernées par des enjeux d'attractivité mais aussi une dégradation financière inquiétante ces derniers mois, l'établissement avait vu sa situation s'aggraver à l'Automne dernier lorsque des fournisseurs avaient fait savoir qu'ils bloquaient les comptes et refusait de livrer les commandes. Au-delà des mesures d'urgence prises. C'était donc une réflexion structurelle qui était nécessaire, portant notamment sur la question du double sites caractéristiques ancienne de l'établissement. Plusieurs pistes ont été étudiés, le 21 février, un conseil d'administration a eu lieu sur site avec des représentants de l'ARS du conseil départemental de délibérations ont été adoptées l'une concernant le transfert des lits du site de cabane vers le site de nos Weiss l'autre concernant le projet d'évolution de l'offre de prise en charge par la transformation d'un pôle d'activité et de soins adaptés de jour en pas à de nuit sur le site de mauvaise et la création d'un centre de ressources territoriales couvrant en priorité la commune de cabane. À ce jour, les résidents du site de cabanes ont disait transférés vers les EPHAD environnants, dont celui de nos en priorité un accompagnement personnalisé de chacun des résidents avec très tôt été mises en place avec nomination d'un psychologue pour faciliter cette orientation. Le personnel titulaire a par ailleurs été entièrement repris par le site de mauvaises. Je sais que l'Agence Régionale de Santé reste pleinement mobilisé sur ce dossier est particulièrement attentive au suivi des conséquences pour la commune de cabane pour les résidents, les familles et les professionnels. Merci madame la ministre et la parole est maintenant à notre collègue Denis Bois-d'. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. La question sert des associations du secteur sanitaire et social. Acteurs de proximité essentiel dans la vie dans nos territoires. À travers leur action en matière d'insertion d'hébergement ou d'accompagnement social. Ces associations réalise un travail indispensable ma faveur des plus fragiles. La qualité de leur travail. Un partenariat étroit avec les élus locaux a d'ailleurs été unanimement salué au moment de la crise Covid. Incite depuis plusieurs années, ce secteur est marqué par la forte expansion de grands groupes, dont le siège se situe bien souvent en zone urbaine. Et dans le Champ d'action s'étend sur l'ensemble du territoire national. Cette transformation du paysage associatif s'explique en grande partie lorsque logique de prestation qui détermine désormais les relations entre les pouvoirs publics et les associations. Depuis plusieurs années, on observe la multiplication des appels à projets et appel à manifestation d'intérêt général. Si ces outils vise un objectif de rationalisation des dépenses publiques que l'on peut partager. On peut néanmoins s'inquiéter de la concurrence générée au détriment des associations intermédiaires fortement implantés sur nos territoires. Cette association et le génère de l'emploi local en développé une réelle expertise sur leur territoire. Elles sont aussi les garante de l'innovation sociale face à la homogénéisation des solutions. J'ajouterai que dans un souci d'efficacité de nos politiques publiques en tout intérêt à préserver le pluralisme associatif à peine de s'assurer une diversité des interlocuteurs. Ma question est dans le simple Madame la Ministre. Compte tenu de son efficacité sur le terrain, notamment dans nos territoires ruraux et périurbains, comptez-vous mettre en oeuvre. Quand comptez-vous mettre à niveau pour préserver notre tissu associatif local rééquilibrer le rapport de force aujourd'hui. Fossé entre les grands groupes et les associations intermédiaires. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur. Vous avez raison de le souligner, le pluralisme de notre ce tissu associatif est une richesse qu'il nous faut préserver au plus près de nos concitoyens, les associations, petites et grandes font preuve d'initiative répondre à des besoins précis accompagnent les publics les plus précaires. Le gouvernement le rend bien sûr hommage et est à leurs côtés en soutien, j'entends vos remarques sur la concentration et la polarisation du secteur qui mériterait d'être objective Je ne tiens pas cependant opposé les petits et les grands qui offre en complémentarité. Le plus souvent dans de très bonnes conditions. Nous avons besoin d'acteurs au réseau développé capables de porter des programmes ambitieux. Nous avons aussi besoin de plus petites structures au niveau local, parfois plus Agile. Un exemple le Ministre des Solidarités de l'elle a de l'agriculture ont lancé il y a un peu le programme. Mieux manger pour tous, doté de 60 millions d'euros en 2023 et qui aura notamment vocation à soutenir les démarches innovantes des territoires. La responsabilité du gouvernement en la matière et de parler à tous les acteurs de tous les soutenir lorsque les difficultés s'accentue. C'est ce que nous avons fait en les accompagnant dans la mise en oeuvre des mesures de revalorisation salariale liées au Ségur, c'est encore ce que nous faisons en cette période d'inflation avec l'application des mesures comme le bouclier tarifaire à toutes les structures. Il nous faudra bien sûr aller plus loin. Vous savez que le secrétariat d'État auprès de la Première ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative mène actuellement des Assises de la simplification associative et donneront lieu à une feuille de route pour mettre en oeuvre des projets précis, les dirigeants et bénévoles des associations de toutes tailles sont associés à toutes les phases de cette concertation, c'est aussi une autre façon de continuer à servir ce pluralisme qui nous est cher. Merci Monsieur Wade. Il vous reste 15 secondes. Madame la Ministre j'entends j'entends votre réponse et je ne suis pas loin de la partager, mais j'attire votre attention sur les difficultés peut que peut connaître, associations de proximité qui sont pas toutes très petite. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Else Joseph. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. L'aide à domicile et l'aide à l'autonomie des personnes sont indispensables dans notre société. Ce sont des missions auxquelles un conseil départemental ne peut se dérober. Il y a quelques mois le département des Ardennes a voté la revalorisation de l'indemnité kilométrique à 45 centimes d'euros pour tous les personnels qui interviennent dans les services d'aide à domicile. Par le département, ceux-ci n'avait pas été fait depuis 2008. Cette revalorisation est essentiel mais nos départements ne peuvent à eux seuls supporter des charges qui ont un impact sur leur budget Pierre témoins de rappeler 1 trop souvent méconnu à Paris 600.000 euros de plus, cela semble dérisoire epsilonesque mais dans les Ardennes. Cela représentait un point de fiscalité lorsqu'on pouvait lever l'impôt, c'est une charge qui conduit à faire des choix. Nous n'avons pas voulu sacrifier l'aide à domicile parce qu'au-delà des chiffres il y a les personnes l'humain, le lien social. des les personnes à domicile, c'est un cri du coeur ne département n'entend pas se dérober à sa vocation de solidarité. Mais c'est aussi un cri d'alarme ne laissait pas nos conseils départementaux seule. La situation est délicate en ce moment infirmière territoriale infirmières libérales et aide à domicile sont mises sous pression et se dépensent sans compter alors que leurs charges sont nombreuses et reconnues leurs conditions de travail se sont dégradées. Ainsi la spécificité des infirmières territoriale mériterait d'être en compte l'accompagnement qu'elles exercent et personnalisée et apprécier leur avis et précieux que ce soit auprès de la commission Mobilité du département ou pour l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées, elle s'implique dans le réseau départemental Madame la Ministre qu'envisagez-vous pour que l'aide à domicile appuyer comment revaloriser ce beau métier d'aide à domicile, comment faire enfin pour qu'il reste attractif et ce à quelques jours de la journée nationale des aides à domicile. Merci, madame la Ministre. Monsieur le président, madame la sénatrice. Conscient des difficultés de recrutement dans les métiers du soin et de l'accompagnement à domicile. Le gouvernement a pris des engagements forts pour développer l'attractivité de ces métiers, notamment en matière de mobilité. Le gouvernement ainsi agréer l'avenant 50 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile qui revalorise le montant des indemnités kilométriques depuis le premier octobre 2022 les salariés relevant de cette branche se voir rembourser leurs frais de déplacement à hauteur de 38 centimes d'euros par kilomètre, contre 35 auparavant. Alors remise sur les prix des carburants qui avaient été mises en oeuvre jusqu'au 31 décembre 1022 a par ailleurs succédé l'indemnité carburant de 100 euros qui a permis de soutenir les travailleurs qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Cette aide a bénéficié aux millions de Français ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14.700 euros notamment un certain nombre d'aide à domicile pour un Français qui parcourt 12.000 kilomètres par an, ce qui correspond à la moyenne nationale. Ces indemnités représentent une aide un peu plus de 10 centimes par litre. En outre, afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques. Le forfait mobilité durable, porté par la loi d'orientation des mobilités offre aux employeurs la possibilité d'attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux salariés privilégiant les modes de transport dits à mobilité douce ce forfait exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 700 euros par an et par salarié en 2022 et 2023, il a été adopté par les partenaires sociaux dans de nombreuses de SMS via des accords collectifs locaux agréée par l'État. Il est également important de rappeler que les conseils départementaux peuvent aussi mettre en place des dispositifs de soutien à la mobilité. Je pense par exemple aux initiatives qui permettent de cofinancer la location ou l'achat d'un véhicule ou la mise en place d'une flotte de véhicules. Bien sûr, il nous faut continuer à réfléchir ensemble dans le cadre d'une démarche plus large d'attractivité aux mesures complémentaires qui pourraient être mises en oeuvre pour soutenir la mobilité des professionnels. Le ministre Jean-Christophe Combe est à ce titre pleinement mobilisée et a fait du sujet de la mobilité des professionnels en point d'intention spécifique du volet bien vieillir du Conseil national de la refondation. Merci pour le 10 secondes. Oui Madame la Ministre j'entends bien vos réponses. Mais je rappelle que nos départements en tout cas le mien est au bord de l'asphyxie et je suis pas convaincu que les réponses que vous venez apporter va améliorer l'attractivité de ce métier. Merci. La la parole pardon et maintenant notre collègue Philippe mouiller. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question, ça porte sur les incidences pour les travailleurs en situation de handicap de l'application du décret numéro 2022 de 57 relatifs au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité. En effet les dispositions contenues dans ce décret ont des conséquences financières injuste et pénalisante pour les travailleurs handicapés et je t'appelle de nouveau le gouvernement. Ce texte introduit une nouvelle méthode de calcul des pensions d'invalidité. Les personnes invalides, dont les revenus d'activité dépasse le seuil du plafond annuel de la Sécurité sociale ont vu le montant de leur pension d'invalidité suspendu depuis septembre 2022 sans qu'elles en soient informés. Ceci entraîne de facto la fin du versement des rentes de prévoyance puisque c'est le otages Getty au versement d'une pension d'invalidité. Les travailleurs handicapés concernés sont donc doublement pénalisés alors qu'ils ont comme les entreprises qui les emploient cotisé pendant des années dans le cadre des contrats de prévoyance. En raison de la perte de leur pension d'invalidité et par conséquent de leurs rentes de prévoyance. Les travailleurs handicapés concernées se retrouve dans une situation financière critique. Certains d'entre eux envisagent même de cesser toute activité professionnelle alors que le travail s'ils n'aiment d'émancipation et d'indépendance financière. Ce texte réglementaire va manifestement à l'encontre de l'esprit de la réforme qui vise à favoriser le cumul emploi-ressources. Si ce texte semble améliorer la situation d'un certain nombre de titulaires de pensions. Nul ne peut toutefois être lésés. Aussi je vous serez reconnaissant de bien vouloir me préciser les mesures urgentes que vous entendez prendre afin de mettre fin à ce, ce qui est vécu par les principaux intéressés comme une véritable injustice et discrimination. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. ou 50% du revenu moyen calculé sur les 10 meilleures années civiles de salaire pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en oeuvre par le décret du 23 février 2022 vice-quant à elle à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaite conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier c'est ainsi 60.000 personnes qui pourront désormais mieux rémunération professionnelle et pension d'invalidité pour poursuivre cet objectif. La réforme a introduit un nouveau seuil de comparaison au salaire antérieur limitée au plafond de la Sécurité sociale, soit 3666 euros brut par mois en 2023. C'est bien sur ce point plus spécifiques que des inquiétudes sont formulées certains assurés dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la Sécurité sociale sont effectivement susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme des mesures effectives rectificatif sont donc envisagées. Sans revenir sur le fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux. Différentes Différentes prestations sociales. Il pourra être relevé pour permettre le maintien des pensions d'invalidité à la grande majorité des perdants actuel de la réforme. Par ailleurs s'agissant des réclamations d'indus de part de certaines caisses primaires d'assurance maladie. Je vous confirme qu'elles sont nulles et non avenues des instructions claires ont été transmises par l'assurance maladie en ce sens, enfin certains assurés disposent une pension complémentaire versée par leur organisme de prévoyance alors même que leurs droits à pension demeurent ouverts certains organismes ont décidé de suspendre le versement avec l'entrée en vigueur de la réforme. Notre analyse juridique confirme que cette suspension ne respecte pas le droit existant et le gouvernement souhaite trouver rapidement une solution concrète. Face à ce désengagement de leur part. Merci. 12 secondes monsieur mouillé. Oui merci Madame la Ministre je vois que vous avez saisies. La difficulté aujourd'hui et que un certain nombre de travailleurs vous proposer un certain nombre de solutions et d'évolution mais il y a urgence puisque depuis septembre 2022, la situation est critique. Voilà donc nous regardons de très près vos propositions. Merci et. La parole est maintenant à notre collègue Daniel Chassain pour la question suivante. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre les accords conclus au terme du Ségur de la santé ont permis des revalorisations de salaires au bénéfice de certaines catégories de personnel, c'est très bien. Malheureusement, nous avons encore des exclus. Depuis le début de la Covid 19. Les employés des établissements médico-sociaux se sont tous mobilisés pour assurer la continuité de service auprès des résidents. Mais depuis l'instauration de la loi Ségur en septembre 2020. Des disparités entre les agents sont encore là hein avec une perception d'incompréhension au sein même de l'établissement pour certaines dispositions bien sûr comme l'obligation vaccinale et c'est normal, ils étaient tous considérés comme des soignants, mais pas pour la prime Ségur en pas ou en centre hospitalier, un cuisinier une lingère un agent d'entretien des locaux, un agent des services techniques, perçoivent le Ségur alors que ces mêmes personnel au sein d'une maison d'accueil spécialisée par exemple l'attendent toujours. Alors qu'ils exercent le même métier, une association qui gère et pas des masses ou dans une masse les faisant fonction d'aide-soignante le secrétariat, les agents d'entretien sont des oubliés alors que dans tous les Ehpad ces mêmes employés. Ont bénéficié de revalorisation salariale. Il est donc très difficile pour les responsables et directeurs, les présidents des conseils d'administration d'expliquer cette situation et il y a des démissions. De nombreuses autres métiers en sont encore exclus. Pour l'instant de dispositifs tels que les techniciens. En radiothérapie ou en radiologie que j'ai rencontrés exerçant en clinique et qui sont au contact des patients toute la journée Madame le Ministre, le gouvernement compte-t-il prendre en considération ces justes revendications élargir l'application des revalorisations salariales prévues dans le cadre du Ségur de la santé. Merci madame la ministre. Monsieur le président, Monsieur le Sénateur, l'attractivité des métiers du secteur sanitaire, sociale et médico-sociale, être au 1er rang de la feuille de route du gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers à ce titre la question de la revalorisation constitue une priorité. L'État aux côtés des départements a pris, d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros. Les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total ce sont près de 700.000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 euros Net mensuels dont 500.000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Lafourcade. Cela concerne notamment les professionnels que vous évoquez qui exerce dans une maison d'accueil spécialisée de la fonction publique hospitalière rattaché à un établissement public de santé ou un Nepad. Suite à la conférence des métiers sociaux de février 2022, le gouvernement a par ailleurs étendu ces revalorisation à 200.000 salariés de la filière socio-éducative exerçant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-, éducatif l'ensemble de ces mesures ont fait l'objet de travaux préparatoires qui ont largement associés à chaque fois les acteurs concernés, association des départements de France, partenaires sociaux, associations des métiers en tension, faisant face à des enjeux d'attractivité importants et nécessitant une action prioritaire de la part des pouvoirs publics bénéficient aujourd'hui d'un réel gain d'attractivité. Pour autant, il convient de poursuivre les actions menées à destination de l'ensemble des professionnels. Le gouvernement est bien conscient que chacun et chacune, contribue à la qualité de l'accompagnement. En ce qui concerne les professions administratif, technique et logistique des autres structures que vous évoquez hors fonction publique territoriale, il convient d'arriver aux côtés des représentants des employeurs et des salariés à la construction d'une convention collective unique pour le secteur social et médico-social. C'est la condition d'une revalorisation durable de l'ensemble des parcours, l'État et les associations des départements de France ont annoncé le 18 février 2022 qu'ils sont prêts à mobiliser 500 millions d'euros pour faire aboutir ces travaux. Les discussions avancent et c'est dans ce cadre que seront traitées les questions relatives à l'augmentation des rémunérations, je vous remercie.

Merci je vais remercier Madame la ministre Agnès Firmin Le Bodo, qui va nous quitter. Après avoir répondu à sa série de questions et accueillir. Madame Olivier Grégoire la ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme pour la série série de questions suivantes. Et je passe la parole à Madame, Laurence Muller-Bronn. Merci monsieur le président, madame la ministre ma question porte sur la diffusion des théories du genre dans les programmes publics et leurs conséquences dans les organismes publics public et leurs conséquences. Voici 2 exemples très concrets. La CAF d'abord a mis en ligne sur son site une campagne intitulée mon enfant et transgenres. Comment bien l'accompagner. Elle affirme ensuite, signe d'une évolution des mentalités, de plus en plus d'enfants et d'adolescents se déclare non binaire ou d'un autre genre que celui assigné à leur naissance cette communication s'appuie sur de larges citations d'associations militantes sans nuance ni avis contraire. Or, non seulement il n'appartient pas à la CAF de définir et encore moins de banaliser un tel sujet mais de plus, ces propos manquent au respect des principes de neutralité et d'objectivité et d'impartialité du service public et surtout en diffusant des contenus qui induisent en erreur les familles, les ministères de tutelle porte une responsabilité sur les conséquences éventuelles de tels discours. À ce propos le ministre de la Santé a été alerté par une tribune signée par des médecins, professionnels de santé et universitaire, lui demandant de faire retirer sans délai cette page pour les raisons que je viens d'évoquer, il proposait également dit réfléchir avec des spécialistes qui alertent les familles sur les manipulations mentales dont sont victimes les adolescents notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui cette page existe toujours le contenu a été modifié à la marge. Un 2ème exemple c'est le planning familial avec le slogan au planning on sait que des hommes peuvent aussi être enceinte ou ou encore la définition des règles survenant chez des personnes qui ont un utérus en gommant volontairement le mot femmes on s'éloigne de la mission d'intérêt général pour laquelle l'État finance le planning familial, c'est-à-dire l'information sur la sexualité et la défense des droits des femmes. Ma question est donc celle-ci, quelles sont les mesures que vous envisagez pour faire respecter le principe de neutralité et d'objectivité dans les campagnes d'information de ces organismes. Merci. Merci, madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Ces dernières années même si votre question. Le le je suppose. Le regard médical et sociétal sur la transidentité, a néanmoins quand même évolué. En 2010, la France, vous le savez a retiré la transidentité de la liste des maladies mentales c'est dire d'où nous partons en réalité. L'OMS a retiré le sujet de la transidentité du Champ de la psychiatrie en 2019. En 2012, le droit français a pu les discours de haine. En 2016, la modification de la mention du sexe à l'état civil a été des médicalisée. Des plans d'action gouvernementaux successifs ont été menées contre les haines et les discriminations anti-LGBT ma collègue, Isabelle Rome, a d'ailleurs lancé le 25 janvier dernier. Les travaux du prochain plan en lien avec l'ensemble des ministères. On estime entre 20 et 60.000 personnes transe genre les personnes trans sont évidemment évidemment ça m'étonne même de devoir le dire mais ça va mieux en le disant des personnes. Qui sont totalement citoyennes, citoyens à part en terre, protégés par le droit français, européen et international. Cette protection juridique octroyées par la France comme de nombreux autres pays s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de juillet 2002. Il s'agit en 1er lieu d'accueillir sans préjugés ni aucun stéréotype les questionnements d'identité de genre et de permettent surtout à ceux qui souhaitent. S'engager dans cette démarche de le faire à cet effet la CAF dans son travail de prévention. à disposition de l'ensemble de la population française. Les informations nécessaires pour assurer l'accès et l'effectivité des droits pour tous les informations élémentaires indiqué sur le site de la CAF ont vocation à rester totalement accessibles de manière universelle. Le débat d'idées ne peut pas se faire au détriment de l'effectivité de droit déjà voté au profit des Françaises et des Français, quel que soit leur orientation sexuelle ou identités de genre. Nous maintenons notre vigilance absolue à commencer par Isabelle Rome et je vous remercie. À titre personnel de cette question. Merci et. La parole est maintenant à notre collègue Christian Klinger. Des Comptes publics. Selon la Cour des comptes, les fraudes sociales détectées coûterait plus d'un milliard d'euros. Je n'ose imaginer le montant réel. Les cartes Vitale actives sont plus nombreuses que les bénéficiaires identifier. Les fraudes liées à la pension retraite suite à la non non déclaration d'un décès sont nombreuses et n'oublions pas les allocations versées indûment. À ces fraudes individuelles jetons les pratiques d'escroquerie sophistiqués et répandus qui rendent ces dernières pratiques difficile à détecter. L'ensemble de ces fraudes témoigne de la gravité des failles de notre système social. Selon la Cour des comptes, les organismes sociaux lutte mal contre ce type de fraude. La cour a ainsi demandé au gouvernement de faire aboutir en 2022. Le recoupement automatisé des fichiers des organismes sociaux à ceux à ceux du Fisc. Depuis 2018, ce rapprochement ne cesse d'être repoussé en mai dernier, le gouvernement indiquait que ce rapprochement serait effectif à la fin de l'année 2022. Aujourd'hui je vous demande où en sont les organismes sociaux dans le rapprochement systématique des coordonnées bancaires utilisés avec celles du Fichier national des comptes bancaires et assimilés appelé Ficoba. Et finalement quand allez-vous mettre enfin en place ces procédures automatisées. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Le réseau des Urssaf a plus que doublé le montant des redressements réalisés depuis 10 ans pour atteindre quasiment 800 millions d'euros en 2022, ça a progressé de plus 46% côté Urssaf depuis 2017. Concernant les fraudes aux prestations et notamment les CAF, les CAF ont détecté 351 millions de préjudice en 2022 soit un triplement en 10 ans et une progression de plus 21% des de de la détection des fraudes depuis 2017. Le gouvernement a donné une nouvelle impulsion. Vous le savez à la politique de lutte contre la fraude sociale dans une feuille de route et un plan d'action annoncée en février 2021, là aussi quelques progrès. Je partage avec vous, même si je connais. Votre mobilisation sur le sujet des cartes vitales et ça n'est certainement pas suffisant mais voici quelques chiffres déjà entre 2019 et 22. L'assurance maladie a procédé la résorption quasi complète du stock excédentaire sur les cartes vitales surnuméraires qui est passé de 600.000 à un peu moins de 3000 réduisant ainsi les risques d'utilisation frauduleuse par ailleurs la fermeture des droits à la protection universelle maladie a été accélérée pour les assurés ne satisfaisant plus aux conditions de résidence stable et régulière. Le renforcement de la maîtrise du risque de non déclaration du décès pour les retraités qui réside à l'étranger et enfin la reprise et la finalisation des travaux de rapprochement automatisé que vous mentionniez, monsieur le sénateur des coordonnées bancaires déclarés en ligne avec le fichier des comptes bancaires dont le déploiement s'effectue progressivement à l'ensemble de la sphère sociale sur surtout 2023 c'est donc tout au long de l'année face à l'évolution et à l'émergence que vous avez mentionné monsieur le sénateur Klinger de nouvelles formes de fraude, un nouveau paquet de mesures législatives a été adopté en loi de financement de la Sécurité sociale ont pour 2023 pour élargir le Champ des échanges d'informations. J'ai peu de temps pour détailler un rendez vous à vous donner une autre action sera menée par le ministre des Comptes publics en vue du PLF 2024 et je ne doute pas que vous serez force de proposition, puisque le ministre Atal s'est engagée encore sur un autre plan de renforcement de lutte contre les fraudes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre Monsieur Klinger vous avez encore. Le temps d'une réplique. J'ai bien entendu votre réponse donc si j'ai bien compris, c'est en 2023 que le déploiement se fera sur le croisement des fichiers, c'est la meilleure méthode et c'est la méthode la plus sain pour détecter évidemment les fraudes importantes et surtout entre départements où par exemple sur le RSA. Il y a quand même quelques professionnels qui qui agissent et qui. M'a qui perçoivent indûment des allocations de nos organismes sociaux donc. On surveillera évidemment cela de près. Merci la parole maintenant à notre collègue Yan Chantrel. Merci. Me. Monsieur le Président Madame la Ministre j'ai été saisi par plusieurs conseillers et conseillères élu des Français de Belgique sur la question de la double imposition que subissent les fonctionnaires binationaux franco-belge travaillant pour l'État français. L'article 10 alinéa 2 1 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, modifié par plusieurs avenants pose le principe que les fonctionnaires français employé en Belgique par l'État français sont imposables en France on a aussi l'année l'alinéa 3 du dit article qui pose également le principe que les ressortissants belges employé en Belgique par l'État français sont redevables de leur impôt en Belgique. Afin d'éviter une double imposition des fonctionnaires. Franco-belge. Notre pays, la Belgique, on est costaud négocié sous couvert de la procédure d'une procédure de concertation prévue à l'article 24 de la convention du 10 mars un accord amiable publié aux militaires belges du 9 novembre 2009 stipulant que les rémunérations exclus du Champ de l'article 10 en application de l'article 10,3 ne sont imposables que dans l'état de résidence du bénéficiaire. Or, dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation de Belgique a considéré que la corde à meubles de 2009 était dépourvu de force obligatoire et qui luttent tribunaux ne peuvent l'appliquer. Depuis lors, les fonctionnaires binationaux franco-belge percevant des rémunérations de sources publiques qui ont été imposées sur leur revenu par la France se voit également délivré des avis d'imposition par les autorités fiscales belges. Cette situation de double imposition de binationaux ayant déjà payé leurs impôts en France a plongé des familles dans des situations personnelles dramatiques avec des montants réclamés pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Le 9 novembre. Il y a une nouvelle convention fiscale qui a été signé à Bruxelles entre nos deux pays, pour éliminer justement les situations de double imposition. Donc, cette convention doit permettre de régler ces ces situations de double imposition. Pour pourtant elle n'a toujours pas été ratifié le nombre de cas de double imposition ne cessent de se multiplier. C'est pourquoi je vous demande les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas encore déposé de projet de loi d'approbation est également pouvez-vous également donné des précisions sur le dialogue engagé avec les autorités belges pour qu'elle prenne des mesures immédiates de suspension du recouvrement des sommes requises et pouvez-vous également assuré que les autorités belges rembourseront bien les sommes perçues par les services Moscou merci. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président toujours hein. Un défi de répondre à autant de questions mais je vais essayer d'aller droit au but. Monsieur le sénateur Chantrel. Vous vous m'autoriserez à passer les formules de politesse pour aller vous apporter des réponses très précises. 9 novembre 2021, la France, la Belgique ont signé la nouvelle convention fiscale sur l'impôt sur le revenu et sur la fortune qui remplace celle de 1964, comme toutes conventions fiscales bilatérales et les chemises au Parlement pour ratification conformément à l'article 53 de notre constitution. Comme vous le soulignez, cette nouvelle convention, elle va clarifier une fois pour toutes le traitement fiscal des rémunérations de sources publiques. Elles reposent sauf exceptions. Sur le principe de l'imposition par l'État qui verse revenus ce principe est logique car ses revenus publics sont financé par les ressources publiques notamment fiscales de cet État. La rédaction de cette clause qui est conforme au modèle de l'OCDE se retrouve couramment dans notre et vos réseaux conventionnels et en particulier dans les conventions négociées récemment. Parallèlement, la Cour de cassation belge a jugé que l'accord amiable de 2008 qui visait justement à clarifier les dispositions de la convention de 1964 relatives à l'imposition des rémunérations de sources publiques pour les binationaux des 2 États était contraire à la Convention encore en vigueur. Elle a donc invalidé entraînant pour certains de nos compatriotes. Une situation de double imposition de leurs revenus. Cette situation insatisfaisante, a donné lieu à des échanges très approfondie et très constructif avec la Belgique, l'intérêt partagé des 2 pays. Hé bien évidemment d'éviter cette double imposition des binationaux. Et donc je profite de votre question, d'abord pour inviter tous les Français qui sont dans la situation que vous décrivez. je vous remercie d'avoir posé la question à se rapprocher du service juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques qui a monté une cellule spécifique dédié qui fera le lien directement avec les autorités belges et je vous confirme sénateur Chantrel, que le gouvernement fait tous ses efforts pour proposer la nouvelle convention à ratification du Parlement dans des délais les plus proches possibles. Je vous remercie. Merci madame la ministre et la parole est maintenant à notre collègue Pierre Jean Verzeaux laine. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur le sujet de la fibre optique. Alors pas sur son enjeu et son utilité, encore plus de pluie depuis le télétravail. Non, ça porte sur le déploiement du réseau de la fibre optique. Je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est celui du département de laine mais qui visiblement se duplique dans pas mal d'autres départements, il y a 10 ans. Est ouvert un appel à manifestation d'intentions d'investissements pour le déploiement de la fibre. En tout cas dans notre département. Les grands opérateurs répondent en l'occurrence c'est Orange et qui fait le choix de dire je vais fibré 2 agglomération Saint-Quentin Laon est une ville, Soissons. Et puis le reste du territoire, la ruralité s'organise. Un syndicat d'électricité prend la compétence de déploiement de la fibre. On est dans ce qu'on appelle les les 10 ans après, c'est un succès sur les RIP le déploiement public il y a 757 communes de fibrer, plus de 220 prise la quasi intégralité du monde rural a été fibré et gratuitement le problème reste finalement dans ce qu'on appelle les zones amis qui sont déployés par les privés. Il y a des engagements qui avaient été pris par Orange mais dans d'autres territoires par d'autres opérateurs et qui ont maintenant l'obligation de fibrer jusqu'à 100 pour % des foyers et nous sommes loin du compte et beaucoup d'habitants et même d'entreprise qui sollicitent l'opérateur leur répond ben non on ne peut pas ou on verra plus tard. Et là il y a pourtant des engagements qui ont été pris. L'Arcep a la possibilité. Soit d'appliquer des pénalités financières, soit de suspendre. La capacité aux opérateurs de pouvoir fournir le le le réseau. Enfin, le but est pas d'en arriver jusque là. En tout cas le cadre il existe et je voulais savoir ce que le gouvernement compte faire le tordre le bras ou tout du moins faire en sorte que les opérateurs tiennent les engagements qui ont été pris, il l'envoi d'une question d'égalité, de justice sur un sujet éminemment important dans l'aménagement du territoire. Merci de votre réponse. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Vert Eulen en juillet 2018, le gouvernement a accepté par arrêté après avis favorable de l'Arcep. Les engagements proposés par Orange. Avec des échéances en 2020 et en 2022 dans votre département, précisément ce sont. ce sont. Que nous allons citer merci. Ce sont pas moins de 59 communes. Qui ont été attribuées à Orange pour en assurer le déploiement. Le gouvernement est conscient des efforts de l'ensemble des acteurs concernés par le déploiement et la réalisation du plan du plan France très, au début des. Et d'autant plus au regard de la crise sanitaire qui a pu ralentir incontestablement les déploiements. Pour autant. Au regard des données chiffrées issu de l'Observatoire de l'autorité de régulation, il est apparu que certains engagements d'Orange n'était juste pas attends. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Sénateur Vert Eulen l'Arcep sur demande du gouvernement a effectivement ouvert une procédure aboutissant à une mise en demeure. Cette décision a été attaqué par l'opérateur. Devant le Conseil d'État qui est en ce moment même en train d'instruire le dossier. Comme vous le savez, la France s'est fixé un objectif ambitieux en matière de généralisation des réseaux en fibre optique à horizon 2025 concernant votre département avec mon collègue, Jean-Noël Barrot. Nous voulons saluer le travail engagé par les collectivités et le conseil départemental qui grâce aux réseaux d'initiative publique a permis de raccorder les 757 communes du territoire et permettre une couverture de 100% fibre. Plus de 95% de vos concitoyens peuvent donc prétendre à un abonnement fibre. Pour autant, Monsieur le Sénateur Vert de laine, vous l'aurez bien compris, vous pouvez compter sur la détermination du gouvernement pour que quand il y a des manquements du côté des des opérateurs l'Arcep saisi. Les les les opérateurs et à son expliquer et à accélérer cette en ce moment même, le cas de l'opérateur que j'ai mentionné, qui a effectué un recours à la suite de la mise en demeure de l'Arcep, demandé par le gouvernement. Je vous remercie. Merci je vais maintenant passer la parole à notre collègue Frédéric Marchand pour la question suivante. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je souhaite évoquer avec vous la situation des salariés des sites des usine Buitoni à Caudry et Théréau Escaudoeuvres. Situés tous 2 dans l'arrondissement de Cambrai, dans le département du Nord. Vous le savez, le site de Caudry a vécu en 2022 des heures sombres suite au scandale des pizzas contaminées à la bactérie E. coli qui a fait une cinquantaine de victimes en France après une fermeture de 8 mois. L'usine a partiellement repris son activité en décembre 2022, le 2 mars dernier. Malgré les efforts déployés par les salariés pour le redémarrage, le groupe Nestlé a annoncé la suspension temporaire de l'activité de l'usine. Il semble à ce jour que Nestlé pour objectif de fermer le site, jetant les 160 salariés et leurs familles dans l'inconnu. Pourtant, le savoir-faire et le sérieux de ceux-ci ne sont plus à démontrer et l'usine de Caudry dispose d'un potentiel industriel performant dans lequel une activité de substitution pour être mises en place dans le même secteur. Autre coup de poignard le j'ai enterré hausse a annoncé la fermeture de la sucrerie décodeur et ses 123 salariés dans le cadre de son projet de réorganisation de son activité industrielle en France, que va devenir la cité du sucre sans sans sucre c'est tout un territoire qui se pose la question et qui est plongé dans le désarroi. La suppression du site des cadavres, a de quoi surprendre puisqu'il se trouve dans une zone de production de betteraves moins touchée que beaucoup d'autre part la jaunisse en 2020. De plus, le marché est porteur et le groupe gagne de l'argent et se désendettent. Cette décision qui a été annoncé de manière brutale est inacceptable. Elle va à l'encontre des engagements pris par terre en 2020 et 2021 sur la pérennité des outils industriels au-delà des 123 salariés cette décision menace en rayon purement et simplement de la carte une sucrerie qui devait célébrer ses 150 ans pour Buitoni et pour la sucrerie cadavres, on retrouve le même schéma, les 2 géants de l'agroalimentaire ont réalisé des millions d'investissements sur les deux sites pour de manière soudaine s'en débarrasser, de manière inattendue, laissant place à l'incompréhension, la colère des salariés, des élus locaux. Monsieur le Ministre de l'Industrie est venu le 13 mars dernier, rencontrer les dirigeants et les salariés des 2 sites à cette occasion, il a été ferme en demandant des comptes aux 2 groupes des garanties pour les salariés et des annonces ont été faites. Madame la Ministre la course contre la montre est désormais engagée et la mobilisation des forces vives du territoire. Mais au-delà de tout le nord de la région des Hauts-de-France et forte pour dénoncer ce coup de force cette brutalité son nom de ces 2 groupes de l'agro-alimentaire, madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer, à ce jour. Quelles sont les avancées du dossier et confirmé la volonté du gouvernement pour venir en aide aux salariés de Nestlé Téréos je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, marchant je commencerai là aussi par la fin et détaillerait mes propos, même si vous maîtrisez parfaitement le dossier. Oui, vous pouvez compter sur l'absolue détermination du gouvernement pour être aux côtés des salariés et aussi pour demander des comptes aux entreprises concernées. Je ne peux pas vous refaire tout le détail vous connaissez fort bien la situation. À à Caudry à Escaudoeuvres. Donc je vous refais pas le constat, vous le connaissez mieux que moi. Vous l'avez mentionné. Mon collègue, le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure s'est déplacé, le 13 mars. Justement pour dire y rencontrer les dirigeants les salariés et surtout, faire le point sur chacune des 2 situations. Étudier les solutions pour les salariés et le territoire à très court terme concernant l'usine Buitoni de Nestlé à Caudry. La direction a annoncé une suspension temporaire de son activité début mars, faute de commandes nécessaires auprès de ses clients. Suite à l'arrêt d'activité, il est aujourd'hui impératif. Qu'une solution soit trouvée par Nestlé pour maintenir les emplois et la production sur le site des réunions de travail entre les services de l'État et les représentants de Nestlé sont en cours en ce moment même pour explorer l'ensemble des solutions possibles. Concernant la situation de l'usine Théréau Saeco d'Oeuvres. Ou d'ailleurs vos, vos collègues députés ont aussi interrogé le gouvernement, de façon totalement légitime. Les explications précises très précises ont été fermement demandé par Roland Lescure à la direction pour justifier cette décision de fermeture. Nous attendons toujours au moment où je vous parle. Leur réponse, il n'est pas admissible pour une entreprise qui a pris des engagements vis-à-vis du gouvernement de ne pas réduire son empreinte industrielle de prendre une telle décision sans en expliquer précisément les raisons économiques, le gouvernement, Monsieur le Sénateur marchand sera aux côtés des salariés du territoire, quel que soit l'issue des deux situations, nous veillerons à ce que chacun des 260 salariés. Une solution et un point de sortie acceptable au sein de leur entreprise ou ailleurs et un plan d'action spécifique sera mis en place pour le territoire. Mais pour le moment, nous attendons des réponses notamment. Sur le site de Théréau ça Saeco d'Oeuvres et je peux vous garantir pour être colocataires à Bercy du ministre-Lescure qu'il n'est pas une heure sans qu'il soit sur ce dossier, je vous remercie. Merci madame la ministre et la parole est maintenant à notre collègue Bernard buis. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre depuis 2022, la Commission européenne a initié le projet de modifier les règles concernant l'étiquetage des modes d'élevage des volailles. Les normes actuellement en vigueur qui existe depuis 1991 autorise l'utilisation exclusive de 5 mentions valorisantes pour l'étiquetage de la viande de volaille. L'objectif étant le suivant, informer le consommateur, de leur mode d'élevage. Une telle réglementation a eu pour effet de créer une segmentation. Il y a un étiquetage clair permettant ainsi aux productions de volaille fermière d'être mieux identifier. Mais le projet présenté par la Commission européenne fin 2022 propose de supprimer l'exclusivité de la liste des cinq mentions valorisantes, risquant ainsi d'entraîner l'apparition d'un grand nombre de mentions incontrôlée. Une telle évolution représente une menace tant pour le modèle agricole français que pour la production de volaille alternative qui plus est dans la région. Auvergne-Rhône-Alpes 4ème bassins de production de volailles de France regroupant environ 2500 éleveurs ou plus de 50% des surfaces de bâtiment de production avicole sont dédiés aux filières fermière. Je pense notamment au Label rouge et au bio. Alertés par des élus locaux et des acteurs professionnels du secteur. Je tenais donc à interroger le gouvernement pour connaître sa position sur un tel projet de révision des normes manifestement contraire aux objectifs visant à soutenir la production locale et durable issu du Green Deal européen et de la stratégie de la ferme à la table. Par conséquent, Madame la Ministre que prévoit le gouvernement pour s'opposer à l'évolution, envisagée par la Commission européenne qui risquerait d'engendrer de graves conséquences en matière de préservation de filières d'excellence et de protection des consommateurs. Enfin, pourriez-vous nous préciser dans quel sens les négociations évoluent et quand est-ce qu'une décision finale aboutira. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Buy une réforme a été initié par la Commission européenne au cours de l'année 2022 sur cette question précise des normes de commercialisation. Le projet de texte transmis en janvier aux États membres a suscité beaucoup beaucoup beaucoup d'inquiétude. De la part des professionnels sur 2 points. D'abord, l'obligation d'étiqueter tout de viande de canard ou d'oie issu de la production de foie gras avec la mention issus de foie gras et d'autre part une dérégulation de l'usage des mentions valorisantes pour l'étiquetage de la viande de volaille jusqu'alors limitée à une liste fermée de 5 mentions valorisantes. Les évolutions qui était initialement envisagée aurait pour effet de décupler les risques de concurrence déloyale entre opérateurs et de décupler aussi les risques de tromperie des consommateurs. Sujet qui m'interpelle particulièrement puisque j'ai aussi l'honneur de m'occuper de la consommation. On est donc bien conscient que ces normes revêtent un intérêt majeur au plan économique pour la filière volaille française. La France a engagé un gros travail auprès de la Commission européenne, pour préserver les intérêts de nos filières d'excellence et garantir la visibilité nécessaire aux productions de volailles extensive en plein air. Le travail porte ses fruits aujourd'hui puisque la Commission européenne a soumis à l'avis des États membres. Un projet de texte qui satisfait plus en tout cas les professionnels avec d'une part le retrait de l'obligation d'étiquetage des viandes avec la mention issus de foie gras et d'autre part une rédaction d'un compromis qui protège et maintient surtout l'exclusivité de l'utilisation des mentions plein air. Soyez assuré, Monsieur le Sénateur Buy que la France malgré ses a enfin en plus de ces avancées continuent à être mobilisés sur ce projet de texte qui doit encore passer plusieurs étapes avant sa publication finale d'ici quelques semaines, je vous remercie. Merci madame la ministre et je vais maintenant passer la parole à notre collègue Mathieu Darnaud pour la question suivante. En Ardèche, comme ailleurs chanteront nous encore le temps des cerises. Au moment où les 855 hectares de cerisier ardéchois s'apprête à fleurir les arboriculteurs se sentent désarmés pour faire face. Aux drosophile Suzuki ce moucheron qui peut détruire, de 30 à 100% des récoltes en effet après l'interdiction du diméthoate en 2016 la Commission européenne a dans son règlement d'exécution du 24 janvier 2022. Refusé. De renouveler l'homologation du Faust mètres dont l'efficacité est pourtant reconnue. Or, cette décision intervient à l'heure où les solutions alternatives, notamment à base d'insectes stériles ne sont pas encore opérationnels. Bien sûr il existe des filets anti-insectes mais leur efficacité, comme on a pu le constater en 2022 dans les vergers voisins du Gard reste très limité. De plus ils sont chers et complexes, a installer dans des terrains accidentés comme ceux de notre département de l'Ardèche, madame la Ministre, le gouvernement s'était engagé à ne pas supprimer de produits phytosanitaires tant qu'une alternative efficace n'était pas disponible. Ma question est donc simple, allez-vous agir pour permettre dans le court terme et j'allais dire dans l'urgence de déroger à l'interdiction des molécules telles que le Faust mettent où le diméthoate. Merci, madame la Ministre. Merci monsieur le. Président Monsieur le sénateur d'Arnaud déjà je j'appelle votre indulgence. Je maîtrise moins bien que vous ce sujet et il y a un certain nombre. De. Relatif aux dérogations que je risque d'écorcher donc je m'en excuse par avance. La France n'envisage pas de réautorisation. Des produits à base de diméthoate et de fausses comme vous le savez, compte tenu de la forte toxicité du diméthoate pour les être s'humains les limites maximales de résidus ont été abaissé au minimum analytique. Ils ne sont plus compatibles avec une utilisation avant récolte. Le Faust mettent quant à lui présente des niveaux de toxicité comparables selon les avis scientifiques. Ce qui a justifié de mettre fin à son utilisation au niveau européen. Conscient évidemment des inquiétudes que cela peut engendrer pour certaines filières. Le ministre-Fesneau a chargé le délégué ministériel pour les alternatives aux produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales. De coordonner un groupe de travail qui ceci les principaux acteurs de la filière cerises et de la recherche agronomique. La première priorité de ce groupe de travail et d'ajuster justement la stratégie de lutte contre la Drosophila Suzuki sur les cerises en envisageant une palette de solutions disponibles avec comme boussole qu'elle ne comporte pas de risques. Il avait oeuvré pour la santé humaine.

demandes de dérogation. L'une a déjà été octroyé les 3 autres sont actuellement en cours d'examen. Il faut en parallèle assuré que les produits végétaux mis sur le marché en France, répondent au même niveau d'exigence. Ainsi la France a d'ailleurs à demandé à cet effet que la Commission européenne abaisse sans délai la limite maximale de résidus en fausse mettent sur les cerises pour s'assurer que les cerises importées en 2023. Depuis cet être traités avec cette Le ministre de l'Agriculture a indiqué à la filière qu'il était prêt à examiner, monsieur le sénateur d'Arnaud. La faisabilité d'un accompagnement financier pour les pertes qu'elle pourrait subir en cas d'attaque sévère de Drosophila Suzuki est à votre disposition, j'ai déjà pris trop de temps mais le ministre-Fesneau est à votre disposition sur ce sujet.

et à trouver des réponses dans l'urgence parce que nous connaissons. Ses, ses limites et ses dates. Depuis 2016 et pour l'heure rien n'est encore opérationnel. Donc vraiment j'implore le gouvernement d'agir rapidement.

Oui je souhaite appeler votre attention sur les obstacles qui s'amoncellent sur nos exploitations agricoles. Fin de la dérogation pour les le nez ou nicotine oui d'interdiction du S se à clore. Nouveau règlement imposé à la filière fruits et légumes. Législation hors sol en matière viticole ou encore signature d'accords de libre-échange portant atteinte. À notre production etc Ce sont les contraintes réglementaires. Franco-française qui viennent saper la compétitivité de nos producteurs. Un simple exemple, seuls 68% des substances actives autorisées et utilisé en Europe peuvent être épandues en France pourquoi résultat, notre pays est l'un des seuls grands pays agricoles, dont les parts de marché recule et dont les importations alimentaires ont doublé depuis 2000. Or ces produits importés sont loin l'aide d'être vertueux. Les autres pays sont nettement moins précautionneux en terme de réglementation sanitaire et laissent leurs agriculteurs lits libres de traitement qui ils sont interdits sur notre sol. Ni notre balance commerciale ni. Notre bilan carbone ne peuvent se réjouir de ces choix. Pour. Tendre vers une. Révèle une réelle souveraineté alimentaire.

qui viennent. Contraindre et pénaliser l'ensemble de notre modèle agricole. Merci Monsieur Détraigne et Madame la Ministre. Pour la réponse. Monsieur le sénateur Détraigne après le sénateur d'Arnaud. Je vais là aussi essayer, même si c'est un défi. De répondre à la question technique que vous posez en matière de surtransposition. Votre question elle contient de nombreux thèmes et dans les 2 minutes qui me sont imparties. Je vais juste rappeler de 3 fait hein. Le nombre total de substances approuvée par l'Union européenne est stable depuis de nombreuses années 453 substances sont concernés. Sur ces 453 substances de 194 relève d'une autorisation de produits mis sur le marché en France qui est l'un des pays les Européens avec le plus de substances autorisées. Seules sept substances ont été interdites au niveau national. 5 néonicotinoïde en 2016 et 2 substances ayant un mode d'action identiques. Depuis, c'est cette interdiction. 4 ont été interdites à l'échelle européenne et une 5ème est interdite en usage extérieur ces chiffres démontrent que l'approche de surtransposition doit être relativisée. En revanche, et vous avez monsieur le sénateur Détraigne parfaitement raison de le souligner. Il y a un enjeu majeur à changer d'approche et de stratégie et c'est tout l'objet de la planification écologique voulue par la Première ministre plusieurs principes guident cette action, une action à l'échelle européenne déjà pour éviter les distorsions de concurrence sur le marché commun. Un soutien à la recherche et à l'innovation pour sortir des impasses et surtout trouver des alternatives viables et opérationnel mais aussi une action par la concertation avec les parties prenantes et. des des des agences publiques des instituts de recherche des entreprises privées du monde agricole pour identifier les impasses et surtout avoir une palette de solutions pour en sortir. Depuis 2017, nous avons posé des fondamentaux avec les loi Egalim avec le principe de réciprocité des normes dans les accords commerciaux avec aussi l'accès à l'eau et la protection face aux effets du changement climatique avec le Varenne, de l'eau. Nous poursuivons donc ses efforts et cette méthodologie en posant un nouveau jalon essentiel pour l'avenir de notre agriculture, grâce au futur pacte et surtout au futur projet de loi d'orientation et d'avenir agricole que portera le ministre-Fesneau dans les prochains mois. Je vous remercie. merci madame la ministre et je, je salue votre présence pour cette série de de questions. Merci madame Olivia Grégoire et puis je j'accueille. La ministre de la culture madame Rima Abdul-Malak pour la question suivante. Qui sera posée par notre collègue Céline Brulin. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre à Rouen comme ailleurs les École nationale supérieure d'architecture se mobilisent en ce moment pour dénoncer des moyens financiers insuffisants des contrats d'enseignants précaires et un personnel administratif en sous-effectif et la création de quelques CDD de remplacement sur des postes administratifs ne suffira pas, je crois à éteindre cette colère. La grande fragilité financière des écoles d'architecture les contraint à multiplier des réponses à des appels à projets, voire à solliciter de plus en plus de fonds privés, ce qui est un problème en soi qui se conjugue au fait qu'elles n'ont ni les personnels administratifs ni l'ingénierie pour mener ce travail a bien la loi de finances pour 2023 a acté un indice de rémunération des enseignants contractuels et vacataires à 410, soit à peine 1500 euros. L'utilisation du 49.3 déjà. Ayant annulé un certain nombre d'amendements que nous avions pu faire ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale qui visait à revaloriser cet indice. Pouvez-vous m'assurer Madame la Ministre que la prochaine loi de finances accédera à la demande des personnels d'un indice à 517 ce qui équivaudrait à un salaire d'environ 2000 euros par ailleurs l'arrêté du 24 avril 2018, ne reconnaît pas l'enseignement des langues étrangères pour l'architecture. Conséquence, les enseignants concernés ne peuvent pas être titularisé ni envisagé d'évolution de carrière. Plus globalement, les moyens alloués par l'État s'élève à 8500 euros par an et par étudiant en architecture, contre 10.500 pour les étudiants de l'université et plus de 15.000 pour ceux des grandes écoles, pourquoi cet pourquoi cet écart. C'est d'autant plus injuste que les écoles d'archi comme celle de Normandie, qui est située à Darnétal sont souvent éloignées des Campus. Ce qui ne facilite pas l'accès des étudiants au service du cross, quelles mesures entendez-vous prendre face à cette crise. En sachant que nous sommes devant des enjeux nouveaux, notamment celui de la transition écologique, dont les écoles vont devoir s'emparer d'ailleurs le ministère de la transition écologique ne devrait-il pas contribuer au financement de cet enseignant cet enseignement aux côtés de ceux de la culture et de l'enseignement supérieur, je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. énormément d'espoir pour l'avenir parce que ce sont eux qui vont penser la ville de demain les les logements de demain. La manière d'habiter le monde demain. Donc on a là un véritable enjeu qui pour moi est très important, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu créer un prix pour valoriser ses projets de transition écologique pour les dernières années. Concernant l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie que vous avez cité, là on a eu un cas très spécifique, ou plusieurs congés maladie, maternité se sont cumulés au service formation et qui ont conduit la direction a repoussé d'une semaine la rentrée du du deuxième semestre on a réussi à trouver une solution pour régler cette situation précise, et d'ailleurs les représentants des personnels de de cette école vont être de nouveau reçu ce vendredi par par mes services. C'est important quand même pour moi de vous rappeler tous les efforts qui ont été fait tout de même depuis 6 ans parce que depuis 2017 il y a eu en matière d'emploi. 111 titularisations d'enseignants contractuels 80 créations de postes rien que pour l'année 2023, ça a été une de mes priorités dans les négociations budgétaires 17 postes supplémentaires et une revalorisation des rémunérations, c'est vraiment acté en matière de crédits de fonctionnement, ils ont augmenté de 7% depuis 2019. Et j'ai ainsi sur les travaux d'investissement aussi qui ont été faits à Bordeaux à Grenoble, à Lille, à Lyon, à Saint-Étienne, 75 millions depuis 2021 de de travaux d'investissement 2023, on en a parlé au moment de présentation de mon budget, j'ai vraiment mis l'accent sur les écoles d'architecture avec une augmentation de 20 120 % qui se répartissent à la fois en fonctionnement et en investissement courant ça permet de rectifier le chiffre que vous avez mentionné la de 8500 euros en fait aujourd'hui la dotation par étudiant elle est évalué à 11.000 euros en moyenne. Je pourrais vous donner les détails du calcul. J'ai bien conscience qu'il reste des questions des inquiétudes qui sont légitimes, je continue le dialogue avec les écoles leurs représentants, et soyez assuré de mon engagement pour chercher encore et toujours des solutions, mais les négociations budgétaires pour 2024 n'ont pas commencé. On aura l'occasion d'en reparler, merci. Merci madame la ministre. D'avoir été présente pour répondre à cette question importante sur les écoles d'architecture on vous laisse repartir. Et on accueille. Madame, Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargé des Anciens combattants et de la mémoire pour les questions suivantes. Et je passe tout de suite la parole à notre collègue Cédric Perrin. le 26 janvier 2022 dans une réponse à une question orale votre prédécesseur rappeler que l'obtention de l'honorariat des réservistes au grade supérieur n'étaient pas de droit depuis un décret du 30 septembre 2019. Ce dispositif repose en effet sur une proposition de l'autorité militaire au ministre en exercice qui doit ensuite fondé sa décision sur des critères précis. Une procédure interarmées s'agit d'éviter que l'attribution de l'honorariat à un grade supérieur, soit possible dans des conditions plus faciles que celle par exemple prévu pour la promotion des militaires d'active, ce serait inéquitable et incompréhensible pour les militaires. à ce jour, ces critères et cette procédure ne sont toujours pas déterminées. En janvier 2022. Votre prédécesseur annoncé une révision prochaine à la lumière des conclusions et les recommandations du groupe de travail constitué des représentants de représentants de l'ensemble des forces armées. Et des formations rattacher cette révision qui semblait imminente étaient déjà annoncé dans une précédente dans l'dans une précédente réponse du gouvernement datée du 13 mai 2021 et évoquait déjà l'existence de ce groupe de travail constitué à la fin de l'année 2020 pour définir les actions qui méritait d'être valorisé. Enfin la semaine dernière j'ai lu dans une réponse du ministre des armées qu'un nouveau groupe de travail sur l'avenir de la réserve militaire avait été mis en place le 21 novembre dernier dans le cadre de la préparation de la loi de programmation militaire, un projet de décret seraient en cours qui pourrait être présenté en Conseil d'État avant la fin du 1er semestre 2023. Je ne doute pas un seul instant de la difficulté que constitue une telle tâche mais voilà désormais 3 ans et demi. Madame le Ministre que nos militaires ayant quitté la réserve opérationnelle patiente. J'ai donc de questions. Pourquoi un nouveau décret jamais évoqué jusqu'à l'aurait-il finalement nécessaire que sont devenus les conclusions du groupe de travail initial, celui qui a précédé le groupe de travail LPM. Quelles sont-elles pour avoir été vraisemblablement balayé par le gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur Perrin. Je vous remercie pour votre question relative à la condition d'accès à l'honorariat au grade supérieur pour les réservistes comme vous le savez les attentes concernant la réserve sont fortes dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire pour donner corps à cette ambition. Le ministère des Armées a mis en place 6 groupes de travail, dont un est consacré à l'avenir de la réserve militaire. Comme vous l'avez dit dans dans votre question dans un esprit de coconstruction de cette LPM avec le Parlement. Ce groupe de travail lancé le 21 novembre 2022 à examiner les les mesures susceptibles de rendre plus attractif un engagement dans la réserve. Parmi les mesures concrètes étudiées est issu des travaux préalables. Le sujet de la modification des dispositions réglementaires relatives à l'attribution de l'honorariat du grade immédiatement supérieur aux réservistes fait actuellement l'objet d'un projet de décret cohérent avec les dispositions relatives à la réserve militaire prévus par la LPM ce projet qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique. De la fonction militaire. Pardonnez-moi, à l'été 2022 est actuellement soumis à la consultation interministérielle. Ils devraient pouvoir être présenté en Conseil d'État avant la fin du 1er semestre 2023. Je vous remercie. Merci madame la ministre et je passe tout de suite la parole à notre collègue Philippe Bonnecarrère. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre je souhaiterais tout particulièrement de m'adresser. À Madame, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au sein du monde universitaire attirer son attention sur les établissements qui ne dispose pas de ce qu'on appelle les responsabilités compétences élargies en jargon administratif, Les RC très concrètement. Parmi ces établissements, l'Institut national universitaire Champollion qui couvre note à Albi, notamment le Tarn et l'Aveyron et le 2ème. Établissement Établissement en France le plus sous-encadrés dans sa catégorie, qui sont les établissements dits pluridisciplinaire. Or, santé. Il a pu arriver qu'il y ait des mesures de rattrapage qui soit a pris avec. Des annonces par exemple pour des emplois sur la filière Staps. Ou avec des compléments financiers sauf que, sauf que pour un établissement comme Champollion. Le fait d'allouer nationalement des emplois supplémentaires dont un emploi par exemple pour Champollion ne se traduit pas dans la réalité, dans la mesure où n'étant pas une établissement dit à responsabilité compétences élargies. Ils dépendent d'un plafond d'emplois pour faire bref, aide aux établissements. Vous avez un nombre d'emplois supplémentaires et on dit l'établissement pour lequel on flèche en emploi, mon cher ami, vous avez un plafond d'emplois on ne bouge pas. La décision d'adjoindre des moyens humains n'est donc plafonné ne peut avoir d'effet. Voilà le sens de ma question, madame le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Bonnecarrere. Le pilotage des moyens et des employes des établissements ne bénéficiant pas de RCE fait l'objet d'un examen particulièrement attentif de la part des services. Les échanges avec ces établissements se sont renforcées depuis 3 ans suite à la mise en place d'un dialogue stratégique et de gestion. Il nous a permis d'établir un constat partagé de la situation des établissements de leur contrainte et éventuellement de leurs besoins complémentaires. Linux Champollion qui participent à ces dialogues et l'objet d'un effort significatif financier depuis 2017. Il a ainsi bénéficié de 5, 6 millions d'euros supplémentaires pour les dépenses personnelles de et de fonctionnement sa subvention pour charges de service publié à augmenter. Pas pardon public a augmenté de 2,2 millions d'euros en six ans, soit une hausse de 40%. Ainsi, contrairement à ce que vous indiquez Monsieur le sénateur, le financement d'un emploi stable supplémentaire s'est traduit par un relèvement du plafond, l'établissement a été informé en novembre 2022 par ailleurs un soutien financier complémentaire à louer des 2022 pour la création de 4 emplois supplémentaires s'est matérialisée par une nouvelle augmentation du plafond de 4 ETPT. Notification initiale de 2023. S'agissant du titre de les crédits. Ont augmenté de 2,2 millions d'euros en 6 ans pour prendre rencontrent des revalorisations et l'évolution du plafond d'emplois. Le ministère assure un suivi enfin des consommations des emplois sur le titre de pour éviter notamment un abattement de plafond d'emplois en loi de finances qui résulterait d'une vacance sous plafond supérieur 1%. Le rehaussement du plafond du titre de ne peut pas être automatique. Il est soumis au constat préalables de la saturation de son plafond d'emplois. Je vous remercie. Merci monsieur Bonnecarrere. des sous-dotées de France et je vous invite vraiment à donner corps à une négociation pluriannuelle ainsi qu'un vrai dialogue. Annuel cette fois-ci avec chacun des établissements. Merci et. La parole est maintenant à notre collègue Frédérique Puissat. merci, madame la Ministre, donc ma question porte sur l'absence d'un statut pour les administrateurs ad hoc. Vous le savez, depuis que le décret de parution de cette. Fonction a été créée en 1999, aucun texte n'est venu véritablement encadrer cette profession alors que le son Champ d'intervention ne cesse de grossir au fur et à mesure des, des textes que l'on qu'on a pu voter, y compris dans cet hémicycle, contrairement aux autres mandataires et je pense notamment aux tuteurs et au curateurs rien n'encadre véritablement ce statut en l'occurrence, absence de formation obligatoire. Absence de déontologie des contours de missions qui sont parfois floues, un exercice qui est hétérogène des mandats sur le territoire national et une indemnisation qui est dérisoire au regard du travail accompli. Je sais qu'il avait eu un certain nombre de propositions de loi qui avait été fait à l'époque par un certain nombre de nos collègues députés, ma question est donc la suivante, est-ce qu'il y a.

Merci monsieur le président, madame la sénatrice, plus la sénatrice plus ah pardon je vous remercie pour votre question relative au statut de l'administrateur ad-hoc. Je vous prierai discuter l'absence du garde des Sceaux Ministre de la justice qui n'a pu être présent monsieur le garde des Sceaux partage avec vous. Le constat de ce que l'administrateur ad-hoc ce parrain judiciaire est un acteur clé dans le parcours d'accompagnement du mineur, victime d'une procédure pénale. Un administrateur ad hoc est nommé en cas de conflit d'intérêts ou de vacances dans la représentation des intérêts du mineur dans un procès. La modalité de sa désignation et de son intervention en justice sont prévus aux articles R. 53 et suivants du code de procédure pénale. Le nombre d'interventions des administrateurs ad hoc et d'environ 5 à 6000 par an. Son recrutement doit être plus rapide pour lui permettre d'intervenir au plus tôt le plus tôt possible dans l'intérêt du mineur accompagné sa désignation doit être plus souple, confiée au procureur de la République et non pas comme actuellement à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel. Sa compétence doit être assurée et vérifier notamment par la, par le suivi d'une formation de qualité sur les enjeux de la procédure judiciaire et en terme de protection des mineurs. La mission de l'administrateur ad-hoc mérite d'être. Dans son contenu doit être aussi mieux contrôler pour permettre un véritable accompagnement du mineur dans tous les actes de la procédure dans l'enquête pénale dans les auditions devant le juge d'instruction à l'audience. La tarification des missions est à repenser la revalorisation de la rémunération pour les missions confiées est essentiel. Monsieur le garde des Sceaux annonce à madame la sénatrice, que ses services ont effectivement mobilisés sur ces questions et vont très prochainement pouvoir lui présenter les travaux qui vont permettre la création d'un véritable statut pour les administrateurs ad hoc. Je vous remercie. Merci à la la Ministre de cette intervention qui me rassure. Elle me rassure d'autant plus que un certain nombre de de ces. Professionnels sont regroupés sous forme associative et parfois avec des carences hein de bénévoles qui qui n'arrivent plus effectivement les gérer mais surtout je pense que. compte tenu du fait qu'on a de plus en plus de de travaux qui sont de plus en plus important. On arrive finalement à avoir des recrutements qui peuvent parfois être du recrutement léger et surtout on a une application du droit en France qui n'est pas une application hétérogènes. qui peut poser un certain nombre de difficultés. Donc on suivra avec attention. Les travaux qui seront conduits par le garde des Sceaux, pensez bien interpeller les professionnels de terrain. Je pense qu'ils ont matière à à pouvoir vous répondre et dans l'Isère en particulier, nous avons une association qui est très construit et qui a effectivement un degré de maturité qui à mon avis nécessiterait peut-être que le garde des Sceaux puissent les les consultiez pour pouvoir effectivement affiner ses travaux. Merci beaucoup en tout cas. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Brigitte Lherbier. Monsieur le président, madame ministre, j'aimerais attirer votre attention sur la longueur des délais de justice pour obtenir une audience puis une décision. Les tribunaux n'arrive plus à faire face malgré l'engagement des magistrats et des greffiers de l'ensemble du personnel à Lille, le président du tribunal judiciaire s'est inquiété le jour de la rentrée sous la du manque de personnel, il estime que le tribunal est chroniquement. Sous-évalué en prenant compte des des parents en retraite. De nombreux magistrats. C'est le cas dans toutes les branches du droit en matière pénale est mise en cause attendent plusieurs années alors qu'une sanction immédiate et rapide et ce qu'il a de plus important pour les mineurs, les victimes de dommages physiques

des réparations pour obtenir réparation en droit de la construction longueur pour obtenir un jugement longueur pour assurer les décisions judiciaires. Je vous rappelle que 270 ordonnance de placement d'enfants en danger ne sont pas honorés dans le département du Nord. Le rapport du comité des états généraux de la justice de 2022. Affirmer. Qu'il faut rendre justice aux concitoyens. Pourront nous être suffisamment compétents pour accélérer les procédures se les nouveaux recrutés. Seront-ils formés pour éviter les erreurs dues à leur manque d'expérience, toute la chaîne de procédure judiciaire sera-t-elle concernées par ces recrutements, donnez-nous s'il vous plaît. La situation actuelle de la justice sans nous parler de stock mais de dossiers douloureux en attente parce que nous parlementaires Madame nous recevons toutes ces personnes perdues ruinée en souffrance dans nos permanences et je peux vous assurer, c'est extrêmement grave d'entendre tout ce qu'elle nous dise. Merci, madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Lherbier. Nous sommes comme vous particulièrement préoccupé par la question cruciale des délais dans le cadre des états généraux nos concitoyens nous ont dit très clairement que la justice était trop lente. C'est même le principal grief qui en effet à l'institution. C'est pourquoi Londres des nouveaux moyens historiques supplémentaire. Le gouvernement souhaite que nous puissions diviser par 2, les délits les DVD, les moyens de notre justice. C'est l'objectif 1er de la de la politique menée depuis 2 ans par le garde des Sceaux. À ce titre, l'embauche de de 2000 contractuels au sein des juridictions a d'ores et déjà permis une diminution des stocks ou des dossiers et déjà permis. notamment en matière civile. Entre 20 et 28% selon les juridictions et les contentieux mais nous devons faire évidemment plus. C'est pourquoi la logique du plan d'action présenté le 5 janvier dernier par le garde des Sceaux vise à la réduction de ces délais. Ainsi donc 1500 magistrats et 1500 greffiers vont être embauchés pour la justice judiciaire sur le quinquennat, c'est autant que sur les 20 dernières années. Vous en conviendrez cependant que. 30 ans d'abandon budgétaire politique et humaines ne peuvent être réparés en un claquement de doigts. C'est pourquoi la loi de programmation du ministère de la justice qui sera présenté prochainement permettra de pérenniser ces efforts historique sur le temps long. Le le le, au service d'une justice plus rapide, plus efficace et plus proche du du justiciable. En plus des moyens, il y a des enjeux de complexité des procédures, c'est pourquoi la procédure pénale sera simplifié. C'est également la raison pour laquelle le garde des Sceaux a lancé une grande politique de l'amiable si l'objectif 1er de la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges et de permettre aux justiciables de se réapproprier leur procès l'amiable est également un moyen de favoriser les circuits courts et donc de réduire les délais je sais pouvoir compter sur l'engagement du Sénat avec qui le gouvernement de travaille en parfaite Intelligence pour améliorer la justice de notre pays, je vous je Merci madame la ministre et je vais passer maintenant la parole à d'autres collègues Pierre-Antoine Levi. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre depuis 2022 l'installation de chaudières à gaz dans les logements individuels neufs est proscrite au nom d'un objectif louable, la transition écologique. Concernant les logements collectifs. C'est une sert de cette interdiction était initialement fixée à 2024 puis heureusement repoussé à 2025, afin de laisser le temps au développement de mode de chauffage alternatifs. Cependant, plusieurs incertitudes subsistent, notamment sur l'extension de cette interdiction, rénovation des logements. Cette politique d'interdiction radicale suscite des inquiétudes à plusieurs niveaux. Tout d'abord le réseau électrique français sera-t-il capable de compenser dès 2025 la surconsommation électrique engendrée par l'abandon du chauffage au gaz. Les tensions sur le réseau cet hiver et les appels du gouvernement aux Français pour réduire leur consommation laisse planer le doute. Les surcoûts engendrés pour les consommateurs et les bailleurs collectif contraint de se convertir à l'électricité. Seront-ils compensés. Au-delà de ces problématiques importantes des craintes de la filière gaz françaises sont considérables. Car cette réglementation entraînera inévitablement la perte de plusieurs milliers d'emplois et surtout la disparition d'un savoir-faire reconnu. Ne commettons pas la même erreur qu'avec le nucléaire ou l'abandon programmé de la filière a détourné des milliers d'ailleurs d'ingénieurs et de techniciens qui font aujourd'hui cruellement défaut alors que le secteur revient gras suite à la volte-face du président de la République. Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il de mettre en place pour accompagner et soutenir la reconversion de la filière gaz si l'abandon programmé de cette dernière se confirme, je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Lévy je vous remercie évidemment pour votre question je vous prie d'excuser l'absence. De la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Le président de la République a fixé. Des objectifs très ambitieux en matière de transition énergétique. Être le 1er grand pays industriel à se libérer de sa dépendance aux énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Depuis 2022, la réglementation environnementale R 2020 impose le recours à une part importante d'énergies décarbonnées pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les logements neufs. Cette première échéance s'est imposé aux maisons individuelles et et s'étend progressivement au logement collectif en 2000 Vance cinq et dans les bâtiments tertiaires. Son objectif est de poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions. Tout en diminuant leur impact carbone. Il n'y a à ce jour pas d'interdiction d'installer des chaudières à gaz dans les logements existants des solutions compétitives existe, il s'agit par exemple de recourir aux réseaux de chaleur, ainsi qu'aux énergies renouvelables ou de récupérer tels que les pompes à chaleur, la géothermie de surface les systèmes solaires ou la biomasse certaines aides tire déjà les conséquences de cette évolution. Ainsi MaPrimeRénov principale. Aide à la rénovation énergétique des logements ne subventionne plus l'achat de chaudières au fioul ou au gaz. Le recours aux énergies décarbonnées et génération et générateur de nouvelles perspectives perspectives pour les entreprises désireuses de s'engager dans ces solutions d'avenir avec des enjeux importants de formation et de compétences. Le gouvernement est engagé pour améliorer la la transition des filières industrielles du chauffage vers des énergies bas-carbone plusieurs outils des des déployés par l'État il concours le renforcement des aides Oran au raccordement au réseau de chaleur. Le fond de chaleur et le plan géothermie lancée en février 2023, les actions en cours pour développer l'industrie française des pompes à chaleur qui font l'objet d'échanges avec les filles, les filières contribue également. Enfin, s'agissant du biogaz. Cette énergie décarbonée doit être soutenu, nous avons consommé 480 TWh de gaz en 2021 et nous avons actuellement une capacité d'injection dans les réseaux de 10. TWh de biogaz avec un gisement globale de biomasse qui restera limitée réduire notre consommation globale de gaz n'est donc pas incompatibles avec un développement fort du biogaz. Nous devons faire les 2 afin de sortir au plus vite des énergies fossiles. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à notre collègue Mickael Vallet. Merci, monsieur le Président, bonjour madame la ministre ma question porte sur la méthode de détection de norovirus dans les productions qui colle française. La conchyliculture est fréquemment touchées durant les périodes hivernales par des épidémies de norovirus induite par divers font ce dysfonctionnement pardon des stations de traitement des eaux. Les conchyliculteurs ne sont en rien responsables de ces manquements des stations d'épuration, tout en en payant le prix fort par les restrictions de production et de commercialisation, vous le savez votre département d'élection est concerné comme les la. La Charente-Maritime dans lequel se trouve le plus grand bassin ostréicole d'Europe. Au-delà de ce problème c'est la méthode même sur laquelle reposent ces interdictions qui interroge la détection de génome du norovirus dans les coquillages n'informe pas correctement sur l'infectiosité du virus puisque le génome peut rester présent après que le caractère infectieux du virus a fortement décliné. Alors qu'une discussion a lieu actuellement au niveau européen pour l'ajout de critères microbiologiques relatifs au norovirus dans le règlement en se basant notamment sur la détection du génome, je souhaiterais savoir où en est concrètement l'avancée du programme de recherche dis Auxiliaire de que le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient et qui se propose d'estimer le caractère infectieux du du norovirus par l'utilisation d'un indicateur virale externe en l'occurrence, ce qu'on appelle les bactériophages fécaux pour que celui-ci devienne à l'instar de ce que font d'ailleurs, l'Australie et les États-Unis. La norme sur laquelle seront prises les décisions éventuelles d'interdiction de commercialisation des production conchylicole pour le dire autrement, fonder une interdiction de vente sur la présence du norovirus. Sans danger pour le consommateur serait un non-sens car ce qui compte ce sont les bactériophages qui eux peuvent être dangereux et qu'une purification d'une vingtaine de jours pourrait suffire visiblement à éliminer. Il faut être pragmatique et avoir une approche scientifique rationnelle dans l'intérêt des consommateurs, des cons qui dit culteurs et de notre balance commerciale. Peu de temps donc compter sur le soutien du gouvernement dans. Ce chemin. Merci, madame la Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur vallée je vous remercie pour votre question relative aux critères de contrôle des norovirus dans les productions donc je suis aussi concerné puisque vous, vous savez que je je suis de l'Hérault et je vous prie d'excuser l'absence du secrétaire d'État de la de la mer. Hervé Berville l'étude. Oxy vire financé à l'aide du Fonds européen pour les affaires mais maritimes et la pêche cofinancé par l'État et la région Normandie a été lancée pour détecter l'infectiosité des norovirus. L'Ifremer travaille également dessus à la suite des résultats prometteurs. Le programme auxiliaire de a été lancée en 2021 pour confirmer la fiabilité de la méthode. Le gouvernement de travaille sur la réglementation pour que les décisions soient prises au plus près des risques encourus par les consommateurs. La méthode du programme auxiliaire de si elle tient ses promesses pourraient être utilisés et permettrait de cibler les norovirus infectieux et éviter la fermeture injustifiée des sites. L'étude devrait être finalisé d'ici quelques mois et la méthode. Une fois validé au niveau national pourrait être présenté à la Commission européenne. Nous continuons de travailler avec les collectivités pour améliorer leur gestion des eaux qui sont responsables de ces contaminations et accompagner les producteurs lors de de ces crises, je vous remercie pour l'intérêt de cette question. Merci madame la ministre donc cette séance de questions orales est terminée, elle a permis de poser 44 question au gouvernement ce matin. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h 30 pour l'examen de de conventions internationales, la séance est suspendue.